Madame la ministre, mes chers collègues, avant de passer au scrutin, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits

Malgré un semblant de rébellion avec la proposition de loi Maurey-Nègre, la majorité sénatoriale et le Gouvernement sont en fait au diapason. Vous êtes d'accord pour changer le statut de la SNCF, pour casser le statut des cheminots et pour ouvrir à la concurrence les transports ferroviaires sans aucune étude d'impact. groupe a été le seul à voter un amendement de suppression de l'article 1 A, qui transforme la SNCF en une myriade de sociétés anonymes soumises au code du commerce. Ainsi, il n'aura fallu que trois jours à la Haute Assemblée pour mettre fin à quatre-vingts ans de service public ferroviaire, livrant aux appétits privés un secteur d'intérêt général. Pourtant, ni le Président de la République ni le Gouvernement n'ont reçu de mandat populaire pour cela. Le président Macron nous apporte la preuve que, loin d'emmener le pays vers la modernité, il en revient, en réalité, aux très vieilles sirènes libérales. Votre légitimité est extrêmement fragile. Elle est même d'autant plus fragile que le résultat du « vot'action

nous avons voulu débattre sur le fond, combattant pied à pied vos arguments et en étant aussi force de proposition. Nous sommes fiers d'avoir bousculé le scénario par la force de nos interventions et par nos amendements. Nous sommes fiers d'avoir porté au Sénat la voix des cheminots, mais aussi celle des usagers, des citoyens et de tous ceux qui refusent une société dans laquelle l'accès au droit à la mobilité sera différent selon que l'on réside en ville ou à la campagne. Un droit dont l'exercice sera lié, demain, au niveau de rentabilité qui en résultera pour les entreprises auxquelles on confiera sa réalisation.

Aujourd'hui, c'est bien le Gouvernement qui porte la responsabilité morale et politique d'un conflit social majeur. Sur le fond, ce projet de loi est dogmatique et technocratique. Il est déconnecté du quotidien de nos concitoyens et ne traduit qu'une obsession pour un libéralisme exacerbé. Ce texte organise l'arrivée de nouveaux entrants en livrant clef en main les moyens et les savoir-faire de l'opérateur public et des cheminots aux intérêts privés transfert de salariés formés, transfert des matériels roulants et des ateliers de maintenance, filialisation des gares ... Autant de « facilités aux nouveaux entrants de bénéficier de l'investissement conjoint de la SNCF et des autorités organisatrices. C'est une véritable distorsion de concurrence Vous vous entêtez, alors que les expériences européennes sont édifiantes : dégradation du service et du coût pour les usagers et dégradation des conditions de travail en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Suède ... Au final, nous ne savons toujours pas pourquoi il est nécessaire de changer le statut de la SNCF. Pourquoi, au lieu des trois établissements publics, est-il urgent de créer quatre ou cinq sociétés anonymes ? L'Europe ne le demandait pas. Pis, ce changement va entraîner une augmentation des taux d'intérêt du fait de la dégradation des notes des agences de notation liée à la suppression de la garantie illimitée de l'État ... Pour aller au bout de son projet de libéralisation, le Gouvernement est même prêt à à reprendre une partie de la dette à hauteur de 35 milliards d'euros. Vous vous gardez bien, toutefois, d'expliciter à la représentation nationale le scénario envisagé et la structure de la dette reprise, et ce malgré nos multiples interventions. Finalement, il s'agit d'une stricte obligation comptable liée aux règles sur l'endettement des sociétés anonymes. Et c'est cela que vous érigez en symbole de l'engagement de l'État. Soyons clairs il ne s'agit en aucune manière de donner plus de marges de manoeuvre à SNCF Réseau, puisque, dans le même temps, vous avez fait adopter une nouvelle règle d'or qui contraint drastiquement les investissements, notamment dans le réseau secondaire. Le président Macron est en quelque sorte entré dans cette réforme, au nom de l'équité, par la dénonciation du statut des cheminots, jetant ceux-ci à la vindicte populaire, organisant le « tous contre tous ».

La presse du week-end ne tarit pas sur les concessions faites au Sénat. Franchement, nous ne voyons pas de quoi il s'agit puisque tous les principes directeurs ont été confirmés.

Il faut tout de même avoir à l'esprit que nous assistons à une grande première : le transfert de salariés statutaires d'une entreprise publique vers une entreprise privée. Au-delà du profond désaccord sur l'ouverture à la concurrence et le changement de statut de la SNCF, vous avez refusé toutes les assurances que nous proposions en repli : un transfert fondé exclusivement sur le volontariat et un véritable droit de réintégration au statut sans limitation dans le temps. Enfin, moins de trains, puisque c'est à cela que va conduire la concurrence, c'est plus de cars, plus de camions, plus d'avions pour un coût environnemental que nous n'avons pas le luxe de nous payer.

et une réelle priorité au rail. Nous le répétons, cette réforme est avant tout idéologique. Elle montre combien le président des riches et son gouvernement ont décidé de s'attaquer aux citoyens et aux salariés. Après les APL cet hiver et les pseudo-privilèges des cheminots aujourd'hui, viendront demain des aides sociales et les retraites. C'est cela votre projet de société : détruire les acquis sociaux et les garanties collectives en laissant les individus démunis devant la mondialisation capitaliste. La réforme de la SNCF est un symbole, madame la ministre ; c'est un repère social que le Gouvernement et le Président de la République veulent faire sauter. Nous voterons contre ce projet de loi dont nous continuons à demander le retrait. Il va à l'opposé d'une réforme ambitieuse pour construire le service public ferroviaire du XXI siècle, écologiquement responsable et répondant aux besoins de la Nation. Avec ce texte, vous ne préparez pas l'avenir, madame la ministre, vous nous engagez dans une voie de garage.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, dans quelques instants, au terme de vingt-cinq heures de débat, nous aurons à nous prononcer sur un texte très important : le projet de loi portant réforme du système ferroviaire. Dans cette affaire, tout avait pourtant assez mal commencé. Le Premier ministre, sans aucune concertation avec les parlementaires, avait annoncé, le 26 février dernier, que la réforme se ferait par ordonnances. Le Sénat, au premier rang son président, avait alors réagi fermement pour dénoncer cette procédure. Un peu plus de trois mois plus tard, la situation a évolué positivement. Le Gouvernement a accepté de limiter le recours aux ordonnances en introduisant, au fur et à mesure des débats, des dispositions législatives. La ministre des transports a eu l'intelligence de comprendre que le Sénat n'était pas dans une posture politicienne qui le conduirait à s'opposer par principe à ce texte. De ce fait, elle a choisi de travailler avec nous dans un esprit constructif et ouvert pour mener à bien cette réforme. L'Assemblée nationale, pour une fois, n'a pas prétendu tout régler. Et le Sénat, comme toujours, a eu à coeur de privilégier l'intérêt général sur toute autre considération. Il convient, à cet égard, de saluer le travail de la Haute Assemblée et l'implication personnelle et très active de son président, Gérard Larcher.

En commission, tout d'abord, grâce au travail remarquable de notre rapporteur, que je tiens à féliciter et à remercier vivement, puis en séance publique, guidés par quatre objectifs : renforcer le volet « aménagement du territoire » de ce texte ce texte ; offrir aux salariés de réelles garanties en cas de transfert ; poser les conditions nécessaires à la réussite de l'ouverture à la concurrence ; maintenir un haut niveau de sécurité et de sûreté au sein du système ferroviaire.

Or nous savons que le système de modulation des péages proposé par le Gouvernement ne suffira pas à éviter que des dessertes TGV disparaissent au nom de la rentabilité.

Pour garantir la pérennité des dessertes menacées, il faut aller au-delà. Il faut que l'État conclue, si cela s'avère nécessaire, des contrats de service public comme nous l'avions déjà prévu dans notre proposition de loi, adoptée par le Sénat le 29 mars dernier. Nous avons donc réintroduit ce dispositif. Sur le volet social, la commission a complété le texte de l'Assemblée nationale. Le rapporteur et moi-même avons reçu les syndicats et recherché, avec le soutien du président du Sénat, les voies et moyens de lever les inquiétudes légitimes des salariés. Nous avons voulu être pragmatiques et humains. Nous avons donc précisé les conditions du transfert en favorisant le volontariat. Nous avons également proposé un dispositif de retour permettant aux salariés transférés, dans un délai de trois de réintégrer le statut en cas de réembauche par le groupe SNCF. En séance, à l'unanimité et avec le soutien du Gouvernement, nous avons décidé d'aller plus loin et de prolonger ce délai de deux ans. Ce dispositif, qui répond à une préoccupation forte des cheminots, devrait contribuer à rassurer ceux-ci. En ce qui concerne les conditions d'une ouverture réussie à la concurrence, nous avons tenu à conforter l'autonomie de Gares & Connexions en tant que filiale de SNCF Réseau pour préserver ses capacités d'investissement, ce qui est tout à fait essentiel. Nous avons aussi soumis la mise en oeuvre de deux dérogations à l'obligation de mise en concurrence- la dérogation pour circonstances exceptionnelles et la dérogation dite de compétence, deux notions un peu floues -à l'avis conforme de l'ARAFER pour éviter des interprétations excessives et, surtout, pour sécuriser le choix des autorités organisatrices qui souhaitent y avoir recours En matière de sécurité, nous avons voulu renforcer la coordination entre les acteurs en autorisant la création d'un groupement d'intérêt public pour assurer des missions transversales utiles au bon fonctionnement du système ferroviaire. Le texte qui vous est proposé, mes chers collègues, constitue donc, comme l'a dit Mme la ministre, un point équilibre. J'espère que son adoption ainsi que les annonces du Gouvernement sur la dette permettront enfin de sortir d'un conflit social qui n'a que trop duré. Je dois à cet égard me réjouir que le Gouvernement et le Président de la République, malgré la pression des syndicats, n'aient pas fléchi. Je tiens à les en féliciter.

Tous ces amendements, je le répète, ont été rejetés. Toutefois, nous serons particulièrement attentifs à ces questions lors de la réunion de la commission mixte paritaire au cours de laquelle, je le pense, nous pourrons parvenir à un accord, sous réserve que ces points soient pris en compte. Mes chers collègues, sur ce texte, le Sénat a, comme toujours, prouvé son sens des responsabilités et de l'intérêt général. Il a eu à coeur non pas de faire de la politique politicienne, mais d'agir dans le seul souci de l'intérêt général.

À toutes celles et à tous ceux qui s'interrogent parfois sur le rôle du Sénat, dans l'opinion publique ou même au sein des instances gouvernementales, je crois que nous avons apporté une réponse claire et nette. faudra, madame la ministre, que le Gouvernement s'en souvienne lors des discussions à venir sur la révision constitutionnelle : l'exécutif et, surtout, la France ont besoin d'un Parlement fort et responsable pour mener à bien des réformes d'ampleur. L'examen du présent texte l'a confirmé. La parole

chers collègues, nous tous, les 348 sénateurs et sénatrices de France, par notre travail, venons de démontrer que le Sénat, lorsqu'il est pris en considération, est un élément déterminant du bicamérisme et de la démocratie parlementaire. Vive la République, vive le Sénat ! Merci Je tiens à remercier tous ceux qui ont permis ce débat, les membres de la commission, le rapporteur et Mme la ministre. Pour autant, nous sommes loin d'être satisfaits de la version du texte sur laquelle nous serons amenés à nous prononcer dans quelques instants.

Le Président de la République et le Premier ministre avaient annoncé une loi rapide, par ordonnances, et avaient chacun tenu des propos qui n'avaient d'autre but que de stigmatiser et provoquer les cheminots. Résultat des courses : des ordonnances et une grève longue qui dure encore

preuve de la nécessité de respecter les corps intermédiaires. On ne dirige pas la France comme on dirige une start-up. Néanmoins, madame la ministre, je continue de m'interroger sur cette méthode singulière de légiférer au doigt mouillé, c'est-à-dire sans étude d'impact ni avis du Conseil d'État. De nombreuses questions importantes restent en suspens. Qu'en est-il vraiment de l'avenir des petites lignes, de la capacité financière des régions, ou encore de la modulation des péages et de leur impact ? Qu'en est-il de la nouvelle trajectoire financière de la SNCF après l'annonce très récente du désendettement ?

Nous avons précisé les ordonnances, notamment sur les conditions de transfert et sur la réintégration possible chez l'opérateur historique par le biais de notre amendement rectifié, voté à l'unanimité. Mais nous ne savons pour l'instant rien de plus que la tenue d'une réunion tripartite État-patronat-syndicats. Nous sommes en droit d'obtenir des précisions sur le rôle que vous comptez jouer dans ces négociations et sur ce que vous comptez y défendre. Certes, ces trois éléments sont dans votre texte, mais je ne suis toujours pas convaincu

À l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique et de la transition énergétique, c'est insuffisant. Il conviendrait de valoriser les externalités positives du rail pour permettre un report modal. De plus, un pacte ferroviaire digne de ce nom devrait concerner tout le rail. Or que constate-t-on ? Quasiment rien n'est dit sur le fret. Quant aux petites lignes et à l'aménagement du territoire, aux éventuels nouveaux développements, les imprécisions et incertitudes sont nombreuses, ce qui peut nous conduire à douter. Il ne s'agit donc pas d'un nouveau pacte ferroviaire. Par ailleurs, la nouvelle organisation de la SNCF que vous proposez risque, paradoxalement, d'affaiblir celle-ci, notamment en raison de cette règle d'or très stricte qui inquiète quant aux nouveaux projets de développement du rail, ou encore de la transformation en société anonyme qui va renchérir le coût du financement

des petites lignes et des services sur les tronçons moins fréquentés, atténuant ainsi l'effet réseau du rail. Loin d'une opposition et d'une obstruction systématiques, nous avons soutenu de nombreuses idées nouvelles lors de ce débat ce débat : place croissante de l'intermodalité et des mobilités douces dans nos modes de déplacement, rôle des gares dans les territoires et nouvelles interactions à créer avec les collectivités, mise en oeuvre d'un schéma de desserte d'intérêt national validé par le Parlement- garantie d'égalité entre les territoires -, nécessité de mettre plus de démocratie dans la gouvernance SNCF et d'affirmer le rôle du Haut Comité du système de transport ferroviaire, créé en 2014, pour un fonctionnement plus transparent Certaines de ces propositions ont été partiellement reprises par notre assemblée. Chers collègues, ce mardi, nous sommes toujours sous un régime d'ordonnances et le conflit social, très dur, se poursuit.

Pour ce faire, il n'était pas nécessaire de provoquer un tel conflit et d'aboutir à un texte qui n'est pas véritablement le nouveau pacte ferroviaire annoncé. Dans ce contexte aussi incertain, nous ne vous donnerons pas un chèque en blanc pour une destination inconnue et voterons contre ce projet de loi. Il

Rendez-vous est donc pris pour les prochains textes, sur lesquels nous soutiendrons encore des propositions ambitieuses et nouvelles, comme cela a été le cas ces dernières semaines. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la réforme du transport ferroviaire que nous allons voter est une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent l'ouverture à la concurrence, la transformation de la société nationale et la fin de statuts professionnels exorbitants du droit commun. C'est surtout une bonne nouvelle pour tous les Français qui subissent chaque année un peu plus les conséquences du retard à réaliser cette réforme. Mais c'est une défaite cuisante pour ceux qui ont organisé la pire des formes de grève, la grève à répétition destinée à pourrir au maximum et le plus longtemps possible la vie de nos concitoyens ; une défaite pour ceux qui prétendent défendre le service public en cassant, depuis des semaines, ce dernier. Ils prétendent défendre un service public qui marche. Nous savons tous qu'il fonctionne mal. Un réseau à deux vitesses avec, d'un côté, les privilégiés des lignes à grande vitesse et, de l'autre, les roturiers des lignes classiques qui accusent un retard d'investissement Tous les élus de cette assemblée peuvent donner des exemples édifiants de cette décrépitude. Les élus des territoires ruraux comme le mien autant que ceux des banlieues de l'Île-de-France ou des grandes métropoles. Le système est usé jusqu'à la corde et tout le monde le sait. Comme est usé jusqu'à la corde le mythe de l'intouchabilité des structures et des statuts publics, alors que, en France-

absence de soutien populaire, fissure du front syndical, érosion du taux de grévistes, détermination du Gouvernement, soutien du Parlement ... Non, 2018 ne sera pas 1995. Et la litanie de l'appel à la convergence des luttes ne fera pas plus advenir un nouveau Mai 68 que la danse d'un sorcier vaudou n'amène la pluie. Ce n'est pas non plus en annonçant chaque semaine des chiffres concernant le nombre de manifestants plus irréalistes que ces jusqu'au-boutistes parviendront à masquer la dure réalité : la marée populaire était une marée basse. La France insoumise, le PCF, le NPA, des dizaines de groupuscules et en plus la CGT, SUD, la FSU

Ce n'est pas avec un référendum bidon, des urnes en carton trimbalées d'un dépôt à l'autre, des feuilles volantes en guise de listes d'émargement et, à la sortie, un score digne de l'élection de Brejnev au Politburo- comme disait Staline, ce qui compte ce n'est pas le vote, c'est la façon dont on compte les votes ce n'est pas avec cette ultime et dérisoire tentative qu'on fera oublier la réalité de sondages convergents : les deux tiers des Français sont pour la réforme et contre la grève. Pourquoi cela ? Parce qu'après des années d'enfumage sur le thème de la grève par procuration, les Français se posent les vraies questions : pourquoi est-ce dans le secteur public, dont l'une des justifications principales est la continuité, que les grèves, donc l'interruption du service pour les usagers, sont les plus fréquentes ? Pourquoi, pour s'opposer au Gouvernement, ses adversaires ne trouvent-ils pas d'autre solution que de s'en prendre aux usagers ? Les jusqu'au-boutistes déguisés en défenseurs de la veuve et de l'orphelin n'étaient pas uniquement dans la rue. Ils étaient aussi ici. J'ai entendu, avec plus d'amusement que de colère, le discours de certains de ceux qui m'ont précédé à cette tribune. Ils continuent à se réclamer d'une idéologie archi-décédée comme ces personnages de bandes dessinées comme ces personnages de bandes dessinées qui continuent de marcher sans s'apercevoir qu'ils sont déjà au-dessus du vide et qu'ils vont tomber dans le ravin. ( Ils ont parfaitement le droit de s'exprimer. Ils ont parfaitement le droit de s'exprimer. Mais il y a un règlement au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, et ce n'est pas par hasard. Je le dis solennellement devant l'ensemble de nos collègues, monsieur le président présenter dans l'hémicycle déguisé avec des chasubles de cheminots revêtues par-dessus des costumes et des cravates, en brandissant des pancartes, de même que venir à l'Assemblée nationale avec le maillot de l'Olympique d'Haudricourt n'est pas compatible avec la dignité de nos assemblées.

Je voudrais en revanche féliciter ceux grâce auxquels notre assemblée est parvenue à produire un texte équilibré et enrichi. Merci à Mme la ministre d'avoir été à l'écoute de nombreuses propositions du Sénat. Merci à M. le rapporteur, Gérard Cornu, qui a réussi un exercice difficile en permettant de rassembler des positions souvent diverses, afin d'aboutir au texte que nous allons voter aujourd'hui. Permettez-moi de saluer également la détermination d'Alain Fouché, qui a défendu au nom de mon groupe de nombreux amendements, dont plusieurs ont été retenus. Enfin, merci à ceux de nos collègues qui ont bien voulu les cosigner et les voter. Cette réforme aurait sans doute pu aller plus loin, et surtout plus vite. Car il faudra attendre encore plusieurs années pour que le nouveau système soit réellement installé, et l'on peut compter sur les embusqués pour mettre à chaque étape des bâtons dans les roues. Mais je me garderai bien de reprocher sa timidité au premier gouvernement qui aura eu le courage de s'attaquer à l'une des vaches sacrées de l'immobilisme français. Il savait qu'il prenait des risques majeurs. Et l'on peut lui pardonner d'avoir dû faire quelques génuflexions bien-pensantes devant des adversaires d'autant plus menaçants qu'ils sont faibles. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi crée enfin les conditions de la concurrence dans le transport ferroviaire. Il donne enfin la possibilité à la SNCF de se réformer pour aborder cette concurrence dans les meilleures conditions et protège les salariés en encadrant les conditions de leur transfert.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous arrivons aujourd'hui au terme d'une réforme qui s'inscrit au coeur du quotidien des Françaises et des Français et concerne un service public historique, partie intégrante de notre patrimoine. Cette réforme est complexe et sensible. Elle souligne la difficulté de concilier des intérêts et des attentes sinon contradictoires, à tout le moins incompatibles parfois. Je veux parler de ceux des usagers, des cheminots, des territoires, ou encore du marché.

Dans le même temps, le secteur ferroviaire ne peut faire abstraction des mouvements qui animent notre monde, qu'il s'agisse des changements sociétaux, de l'évolution de notre contexte politique - je pense bien évidemment à l'Europe -, ou des transformations de notre environnement qu'il est de notre responsabilité partagée de protéger.

Je crois à l'essor du chemin de fer, dès lors qu'il sait s'adapter à l'évolution des besoins et de la concurrence [ ...] ; je crois à la capacité du secteur public pour mener de telles missions en alliant efficacité économique et progrès social. [ ...] Mais [ ...] une grande entreprise publique est aussi celle qui sait associer son personnel à ses propres progrès.

de l'intérêt d'un bicamérisme équilibré, et signe d'un Sénat en pleine vitalité et jouant complètement son rôle de législateur. Notre assemblée a ainsi su répondre à un certain nombre d'inquiétudes exprimées ces dernières semaines, notamment au travers du mouvement de grève que nous connaissons actuellement. On peut ainsi se féliciter de l'inscription dans le projet de loi de l'incessibilité du capital de la SNCF et de garanties certaines apportées à la protection des cheminots. Je n'en citerai que quelques-unes : réaffirmation du statut particulier des personnels, maintien des conventions et accords collectifs, inscription de garanties en cas de transfert d'activité et encadrement des modalités de rupture du contrat de travail en cas de refus du salarié, notamment en matière de mobilité professionnelle. Certains, dont je fais partie, auraient souhaité aller encore plus loin, en particulier s'agissant des limites régionales de la mobilité. Les débats ne l'ont pas permis, mais le texte n'en constitue pas moins une réelle avancée pour les agents concernés en comparaison de sa version initiale. Fidèle à son ADN, la Haute Assemblée a également renforcé la place des collectivités, tout comme celle des usagers, dans un certain nombre d'instances, y compris au bénéfice des personnes en situation de handicap. Attachés à l'équilibre des pouvoirs, nous avons collectivement entériné sur de nombreux points le rôle prépondérant de l'ARAFER, afin que celle-ci puisse jouer pleinement son rôle de garant et de suivi de la mise en oeuvre comme de l'impact de cette réforme.

Enfin, soucieux de ne pas hypothéquer l'avenir, nous avons établi quelques principes financiers pour sécuriser l'évolution de la dette et assurer la soutenabilité pour les opérateurs de l'évolution des redevances. Soulignons encore l'encadrement des dérogations à la concurrence ou du transfert des matériels roulants, même si mon groupe aurait souhaité aller plus loin dans l'intérêt des régions et ancrer l'égalité territoriale au coeur du texte. Car, madame la ministre, où se placera le curseur de la solidarité nationale ? que le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, propose de financer à hauteur de 50 % les coûts de rénovation de la ligne Abbeville-Le Tréport, l'État va-t-il se réfugier derrière la règle du retour sur investissement calculée par SNCF Réseau ou suivre la collectivité prête à s'engager ? je n'évoquerai pas la ligne Brive-Aurillac ! Que se passera-t-il pour les régions les plus pauvres sans péréquation favorable ? Nous devons, mes chers collègues, rester vigilants à ce qu'on ne crée pas des régions à deux vitesses.

ces contrats contribueront à préserver les dessertes TGV cruciales en matière d'aménagement et de dynamisme des territoires, pour des lignes moins rentables. J'oserai une dernière citation, empruntée à Jules Renard, dont le père a travaillé à la construction de la ligne Laval-Caen

vous le savez tous, le Sénat était très attendu sur cette réforme ferroviaire. Je crois pouvoir dire qu'il a été à la hauteur de l'enjeu, fidèle à son sens du dialogue et de la concertation. Le débat a été de grande qualité, et chacun a pu défendre ses convictions dans le respect et l'écoute de l'autre. La volonté du Gouvernement de présenter un projet de loi d'habilitation à légiférer par ordonnances, tout en promouvant le dialogue social pour introduire au fur et à mesure des dispositions concrètes devant a été mal comprise et a eu le don de mécontenter à la fois les parlementaires et les syndicats. La majorité sénatoriale avait le choix entre deux attitudes soit une opposition stérile au Gouvernement, laissant pourrir le conflit entre celui-ci et les grévistes ; soit une attitude plus responsable, pour sortir par le haut de cette épreuve, pour la France et les Français.

cette situation, nous avons choisi la seconde option parce que c'est l'ADN du Sénat d'agir avec responsabilité, en dépassant les clivages politiques. Je voudrais à cet égard remercier personnellement notre président de groupe, Bruno Retailleau, de sa confiance et de son soutien total. Un climat de confiance réciproque s'est également instauré entre la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et la ministre des transports, Élisabeth Borne, qui a permis une véritable coconstruction de la loi. J'espère, madame la ministre, que votre attitude positive envers le Sénat servira d'exemple à certains de vos collègues du Gouvernement.

Nous avons plus que jamais besoin de la sagesse du Sénat, d'un bicamérisme moderne face aux humeurs et aux tensions.

veillé à supprimer au maximum les ordonnances, en ne conservant que celles qui avaient un caractère purement technique. Nous sommes restés fermes sur le cap, l'ouverture à la concurrence, la fin du statut de cheminot et la transformation juridique de SNCF et de ses deux filiales. Toutes les avancées importantes figurent dans le projet de loi, et je ne doute pas que nous pourrons aboutir à une CMP conclusive sur la base du texte voté par le Sénat. L'aménagement du territoire a été au coeur de nos préoccupations, notamment les petites lignes et les dessertes directes TGV sans correspondance pour des villes moyennes qui auraient pu être menacées dans le contexte d'ouverture à la concurrence.

Il fallait lever les inquiétudes légitimes des salariés du groupe public ferroviaire, dont je tiens à saluer l'engagement pour le développement du transport ferroviaire. Nous avons précisé le cadre du transfert de personnel et renforcé les droits garantis aux salariés transférés, notamment en favorisant le volontariat à l'échelle de la région

Nous avons voulu faire taire les rumeurs injustifiées de privatisation de la SNCF, en inscrivant dans la loi que le capital de la société SNCF et de ses deux filiales serait intégralement détenu par l'État et incessible. Pour conclure, je veux m'adresser aux syndicats et aux grévistes. Le groupe Les Républicains

de toutes les avancées sociales validées par la ministre, j'ai la certitude que le texte ne sera pas dénaturé par la commission mixte paritaire. J'y veillerai personnellement. Comme le disait Maurice Thorez

Comme le disait Maurice Thorez ,il faut savoir arrêter une grève des travaux du Sénat vous en donne une véritable opportunité

En terminant mon intervention le 29 mai dernier, j'évoquais l'injonction lancée par Victor Hugo le 21 juin 1877 à notre assemblée

Le train est parti à l'heure indiquée et, après un parcours que certains pensaient parsemé d'embûches, il est arrivé en gare, sans retard, après un voyage sans doute harassant, mais ô combien passionnant

les mêmes tentent de nous expliquer que le débat n'a été rendu possible que par la pression exercée depuis le début du mouvement social. Et si nous arrêtions, pour une fois, de raisonner de manière aussi manichéenne ? Pourquoi cette réforme n'aurait-elle pas été rendue possible par une seule et même volonté, à savoir l'attachement collectif au service public ferroviaire ? Cette réforme ferroviaire n'est ni une victoire pour les uns ni une défaite pour les autres. C'est d'abord et avant tout la volonté, partagée sur l'ensemble de ces travées, de préserver notre service public ferroviaire à la française en l'armant de la meilleure façon qui soit face à l'ouverture à la concurrence. Notre expression a été diverse et variée. C'est toute la force de la démocratie, empreinte parfois d'outrance et de mauvaise foi, qui a permis à toutes les sensibilités de s'exprimer en toute liberté de ton et de parole. Je qualifiais le débat de passionnant, car tous les sujets de la réforme ont été abordés, grâce au formidable travail préalable effectué par le rapporteur, Gérard Cornu, et par le président de la commission, Hervé Maurey, qui ont mis leur énergie et leurs compétences au service de la réussite de cet exercice collectif. Oui, l'exercice a bel et Sénat et Gouvernement ont travaillé en bonne intelligence, et nous avons particulièrement apprécié, madame la ministre, l'état d'esprit avec lequel vous avez souhaité, d'emblée, appréhender l'examen de ce texte. Nous nous félicitons également du travail de concertation effectué en amont avec celles et ceux qui ont souhaité discuter et échanger. Vous avez, à de nombreuses reprises dans la discussion, évoqué la notion de coconstruction, et c'est bien cette démarche positive que nous retenons aujourd'hui. Nous allons nous prononcer sur un texte équilibré, qui nous permettra de réinventer la réalité du fait ferroviaire dans notre pays. pays. Nous partageons en effet le même constat : notre système ferroviaire est aujourd'hui en bout de course. Nous avons beau nous réfugier derrière tous les argumentaires possibles et imaginables, la vérité est bien celle-ci l'ouverture à la concurrence qui se profile à l'horizon nous donne l'occasion unique de repenser complètement, de refonder notre logiciel ferroviaire, dans un souci d'efficacité, de modernité et de justice sociale. L'efficacité, c'est d'abord et avant tout la qualité du service proposé aux usagers, en remettant les collectivités territoriales au coeur de la mêlée s'agissant des trains conventionnés. Notre discussion et les amendements adoptés font des régions des acteurs incontournables de l'aménagement territorial du ferroviaire, dans le cadre

La vérité est pourtant simple ; l'incessibilité et l'inaliénabilité sont bien les deux mamelles de notre service public ferroviaire et le resteront. Dire le contraire, c'est mentir à nos concitoyens ; c'est mentir aux cheminots Le texte est suffisamment clair. Le moment est donc venu d'en finir avec ces petites polémiques. Forte de cette garantie, notre société nationale a tous les atouts pour se réinventer et se projeter vers l'avenir dans le cadre d'un projet d'entreprise partagé.

en tentant d'opposer les uns aux autres ne me paraît pas digne des enjeux du monde ferroviaire. Vous avez en effet réaffirmé tout au long de la discussion, madame la ministre, la ferme volonté du Gouvernement d'accompagner les négociations entre l'UTP, l'Union des transports publics et ferroviaires, et les organisations syndicales pour l'élaboration de la convention collective de la branche ferroviaire.

cas de transfert, l'unité sociale au sein du groupe, le retour au statut entre la troisième et la huitième année pour un cheminot qui retourne à la SNCF sont autant de mesures significatives qui donnent sens à la réforme. Il est Il est faux de dire que cette réforme se fait au détriment du monde des cheminots. Ce sont eux les acteurs essentiels de notre grand service public ferroviaire, et des engagements forts ont été pris par le Gouvernement et la représentation nationale. Il n'appartient bien sûr à personne de dicter leur conduite aux organisations syndicales, mais il semble que le moment soit désormais venu d'ouvrir une nouvelle page de notre grande histoire ferroviaire et de réconcilier les Français de tous bords et de tous horizons avec le chemin de fer. Vous le savez, nous le savons tous, l'ouverture à la concurrence est une chance dont nous devons nous saisir collectivement. Il convient là aussi de dire les choses sans agiter de chiffons rouges. Je m'en remets sur ce point à notre régulateur, l'ARAFER, et à son excellent rapport sur le sujet : « Lorsque les pays européens ont utilisé l'ouverture à la concurrence comme un instrument visant à relancer le transport ferroviaire de voyageurs, cet instrument a, de manière générale, porté ses fruits et contribué à une amélioration parfois spectaculaire de l'offre, des performances, de la qualité de service et du prix payé par l'usager. » Parce que « là où il y a une volonté il y a un chemin », le groupe La République en marche votera sans hésiter ce texte pour un nouveau pacte ferroviaire. Mes

La séance est suspendue.

l'étape que nous franchissons aujourd'hui est majeure. Nous venons d'engager la transformation de notre système ferroviaire, pour qu'il s'adapte aux besoins et aux attentes de nos concitoyens.

les membres de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et son président, M. Hervé Maurey, qui ont pris en compte les propositions du Gouvernement et les ont complétées. Je souhaite saluer notre travail commun, qui a été très constructif, chacun dans son rôle, partageant le même objectif de faire avancer la réforme.

Pour les raisons que je viens d'évoquer, je suis confiante, car non seulement les grands axes de la réforme ont été confortés, mais la volonté d'aboutir à un accord pour l'avenir du système ferroviaire français est, je le sais, partagée. Mes chers

Il s'agit, pour Christophe Castaner, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, du premier débat, ici, sur l'application des lois, mais je suis certain qu'il répondra avec précision aux questions qui lui seront posées. Le Sénat procède annuellement au contrôle de l'application des lois. C'est un exercice dans lequel notre assemblée a été pionnière, et auquel nous accordons, chacune et chacun, une grande importance

Il a notamment proposé d'inscrire dans notre texte fondamental une obligation pour le Gouvernement de prendre les mesures générales d'application des lois. Je forme le souhait que les débats que nous aurons prochainement sur le projet de loi constitutionnelle puissent participer à faire de la fonction de contrôle du Parlement une véritable priorité, de même rang que la fonction législative. Au cours de l'année parlementaire 2016-2017, qui vit pour la première fois depuis le début de la V République se succéder élections présidentielle, législatives et sénatoriales, nous avons néanmoins voté 48 textes nécessitant 500 mesures d'application. Sans plus attendre, je donne la parole à notre collègue Valérie Létard, qui préside la délégation du Bureau chargée du travail parlementaire, de la législation en commission, des votes et du contrôle. Je la remercie pour la qualité de son rapport d'information sur le bilan de l'application des lois au 31 mars 2018. Monsieur le 2018. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je me réjouis de l'organisation de ce débat sur le bilan annuel de l'application des lois. En effet, nous n'avions pas eu la possibilité de l'organiser l'an dernier, en raison de l'interruption des travaux en juin. Le Sénat a toujours été très vigilant sur la bonne application des lois et, en particulier, sur la publication en temps et en heure des textes réglementaires prévus par le législateur. Comme les années précédentes, ce bilan est le résultat d'un travail minutieux de chaque commission pour les lois relevant de son ressort. Permettez-moi de saluer la qualité du dialogue avec les administrations et le secrétariat général du Gouvernement, témoignant de la volonté commune du Sénat et du Gouvernement d'une bonne application des lois. Ce bilan s'appuie également sur les données statistiques issues de la base APLEG propre au Sénat. Cette base et la méthodologie utilisée permettent une homogénéité de la donnée dans le temps, garante de l'effectivité des comparaisons réalisées par la Haute Assemblée au fil des ans. Ce bilan porte sur l'application des lois promulguées au cours de la session 2016-2017 au 31 mars 2018. Cette date de référence, six mois après la fin de la session concernée, est choisie en raison de l'objectif que s'est fixé le Gouvernement d'une publication des textes d'application dans ce délai. La session 2016-2017 a été atypique. Pour la première fois depuis le début de la V République, se sont succédé au cours d'une même année parlementaire les élections présidentielle, législatives et sénatoriales. Cela a eu des conséquences sur nos travaux.

Cette proportion est en augmentation par rapport à la session précédente. J'ajoute que l'ensemble des projets des lois ont été votés selon cette procédure. des lois votées lors de la session, 21 lois sont d'origine parlementaire, dont 9 d'origine sénatoriale. J'en viens maintenant au taux d'application des lois. Pour la session 2016-2017, 26 lois appelaient des mesures réglementaires d'application, les 22 autres étant d'application directe. Le taux d'application de ces 26 lois s'élève, selon les calculs du Sénat, à 73 %.

Une précision méthodologique est peut-être nécessaire : le taux d'application, qu'il soit calculé par le Sénat ou par le Gouvernement, est compris comme le rapport entre le nombre de mesures prises et le nombre de mesures attendues il ne tient donc pas compte des articles ou des lois n'attendant aucune mesure d'application. Pour la session 2016-2017, ce sont ainsi 384 mesures, sur les 527 attendues, qui ont été prises.

Sur l'ensemble de la législature, ce sont ainsi plus de 3 000 mesures réglementaires d'application qui ont été prises. Ce taux élevé d'application des lois de la XIV législature s'explique notamment par la très forte mobilisation de l'ancien gouvernement dans les derniers jours de son mandat plus de 400 décrets ont été pris aux mois de mars et d'avril 2017 et dans les dix premiers jours de mai 2017, soit juste avant l'élection présidentielle. Par comparaison, sur la même période en 2016, 147 mesures avaient été prises. Le délai moyen de prise des décrets pour les lois votées lors de la session 2016-2017 est en diminution : il est de cinq mois et dix jours, contre six mois et vingt-deux jours pour la session 2015-2016. Toutefois, encore 30 % des décrets pris le sont plus de six mois après la promulgation de la loi, dont 6 % plus d'un an En outre, le délai de prise des décrets d'application est supérieur à celui du vote de la loi selon la procédure accélérée mois et six jours, soit 158,5 jours, sont en moyenne nécessaires pour les décrets d'application, contre 145 jours pour l'adoption de la loi selon la procédure accélérée. On peut ainsi s'interroger sur le recours toujours plus accru à cette procédure accélérée, face à une lenteur supposée de la procédure législative : en définitive, le Gouvernement a besoin d'un délai supérieur pour prendre les textes d'application- et encore, il publie seulement une partie des textes La période de référence comprend également deux lois de la nouvelle législature appelant des mesures d'application : les deux lois de septembre 2017 relatives à la confiance dans la vie politique. L'ensemble des décrets d'application de ces lois ont été pris. En outre, les éléments transmis par M. Marc Guillaume, secrétaire général du Gouvernement, pour les lois votées depuis le 1 octobre 2017 témoignent d'un engagement fort du nouveau gouvernement. À titre d'exemple, il ne reste qu'un décret d'application à prendre pour la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. Il pourrait être pris avant la fin Dans ces conditions, cette loi serait rendue totalement applicable dans un délai de moins de quatre mois. Ce début de XV législature est donc porteur d'espoir, et nous espérons qu'il annonce une prise de mesures d'application plus complète et plus rapide pour cette nouvelle législature.

Les rapports demandés par le Parlement au Gouvernement dans le cadre d'une loi sont aussi trop rarement remis. Au cours de la session 2016-2017, près de 70 rapports au Gouvernement ont été demandés,

Dans ces conditions, il souhaite pouvoir disposer des documents dont le dépôt a été prévu par la loi. Certains rapports sont remis avec un retard important. Dans d'autres cas, sans aucune explication, ces rapports sont prêts, mais ne sont pas transmis. Par ailleurs, certains rapports ne sont pas transmis officiellement au Parlement, au motif qu'ils sont rendus publics. Or le processus de transmission établi permet notamment de garantir une information rapide des parlementaires sur l'existence de ces rapports.

l'argument de la célérité de l'ordonnance comme véhicule normatif est à relativiser. Le délai moyen de prise de l'ordonnance, calculé comme le temps constaté entre la demande d'habilitation

Je rappellerai ici le contrôle qui vient d'être mené, au sein de la commission des affaires économiques, sur la loi du 1 juin 2016 habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour réformer Action logement.

n'est toujours pas installé, plus d'un an après la mise en oeuvre de la réforme, faute d'adoption des décrets relatifs à sa composition et à son fonctionnement. Or cette structure est fondamentale, car elle est censée jouer un rôle de vigie, au regard des orientations et de la distribution de la participation des employeurs à l'effort de construction entre les organismes et entre les territoires. Monsieur le secrétaire d'État, quand le Gouvernement compte-t-il prendre le ou les décrets concernant le comité des partenaires Je terminerai cette présentation en évoquant les propositions en matière d'application des lois émises par le groupe de travail du Sénat mis en place dans la perspective de la révision constitutionnelle. la création d'un nouvel article 37-2 obligeant le Gouvernement à prendre les mesures générales d'application des lois. En outre, sur le modèle de la saisine du Conseil constitutionnel, il est proposé de permettre aux présidents des deux assemblées, ainsi qu'à une soixantaine de députés ou une soixantaine de sénateurs de saisir le Conseil d'État en l'absence de publication des mesures réglementaires d'application d'une loi dans un délai raisonnable. Vous le voyez, monsieur le secrétaire d'État, notre institution est très attachée à l'application effective des lois que nous votons. Merci, Merci, Monsieur le président, madame la présidente Valérie Létard, mesdames, messieurs les présidents de commission, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de m'accueillir pour ce premier exercice annuel, en cette législature, de bilan et de dialogue sur l'application des lois.

Chacun ici le sait, une loi qui ne serait pas appliquée ne produirait pas tous les effets annoncés et attendus. Elle se limiterait à l'intention, à l'incantation. Or nos concitoyens ont aujourd'hui une exigence d'efficience, parfaitement légitime, et vous êtes évidemment dans votre rôle en relayant

à cinq mois et dix jours en 2016-2017, et le maintien à un niveau élevé du taux d'application pour la session 2016-2017, à 75 %. Ces constats positifs s'ajoutent à celui d'un taux d'application élevé des lois votées sous la XIV législature, qui atteint 93,5 % au 22 mai 2018. Je note en outre que les taux d'application des projets et des propositions de loi sont proches : ils s'élèvent respectivement à 95 % et 91 %- c'est un bon indicateur.

pour obliger les cabinets ministériels, et les ministères, à entrer dans cette logique et à travailler d'abord sur l'efficience de l'exécution, avant d'imaginer produire de nouvelles normes. Ces pratiques vont, me semble-t-il, dans le bon sens. Outre l'organisation de réunions interministérielles pour chaque loi nouvelle, le suivi de l'application des lois fait toujours l'objet de communications

nous organiserons en septembre un comité interministériel de l'application des lois, avec le secrétaire général du Gouvernement et l'ensemble des directeurs de cabinet des membres du Gouvernement, pour maintenir la pression.

afin que les rapports au Parlement, qu'il s'agisse des rapports dits « de l'article 67 » ou des rapports demandés par le Parlement, soient remis dans les formes. J'ai entendu votre message. Vous m'avez interpellé, madame la présidente, sur d'autres sujets, qui devraient revenir

l'absence d'application réglementaire de deux mesures en faveur des consommateurs en situation de précarité énergétique. La première a trait à la mise à disposition d'afficheurs déportés, qui permettraient aux consommateurs possédant déjà un compteur communicant de consulter en temps réel leurs données de consommation. Deux arrêtés sont annoncés pour les prochains mois. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous être plus précis sur le calendrier et les modalités de déploiement de ces afficheurs ? plus ponctuelle, mais non moins essentielle pour ses bénéficiaires : elle concerne l'accompagnement des consommateurs aux revenus modestes qui devraient remplacer un équipement en cas de changement de la nature du gaz distribué- tel sera le cas dans le nord de la France. Faute d'avoir pu introduire lui-même une aide pécuniaire dans la loi, le Sénat avait demandé un rapport, que le Gouvernement n'a pas remis au Parlement. Là encore, monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous dire où en est la mission confiée à pas moins de trois corps d'inspection pour étudier les différentes options juridiques et financières et pour définir les contours de cette aide ? Je le redis, le temps presse ! Je n'évoquerai pas ici la loi de juin 2016 réformant Action logement, sinon pour préciser que je partage toutes toutes les interrogations de notre collègue Valérie Létard. Puisque vous nous y invitez, je réitère sa question sur la mise en place des outils de gouvernance, notamment du comité des partenaires du logement social, seul lieu où les élus Pour finir, je tiens à insister sur la défaillance constante dont fait preuve l'administration en matière de remise de rapports. Les chiffres sont éloquents : un tiers des rapports de l'article 67 attendus par notre commission ont été établis

l'article 28 de la loi que vous avez citée. Trois arrêtés devaient être publiés. Ces trois arrêtés sont aujourd'hui rédigés, mais une évaluation du coût du dispositif par le ministère de la transition écologique et solidaire est en cours. C'est sur le fondement de cette évaluation qu'ils seront publiés. Nous allons relancer la demande, pour pouvoir avancer sur ce sujet. Sur l'aide au remplacement d'un équipement en cas de changement de la nature du gaz distribué, vous aviez effectivement demandé un rapport. Ce rapport a été confié à trois corps d'inspection, Ce rapport a été confié à trois corps d'inspection, qui sont en train d'étudier les différentes modalités, explorant les options juridiques et financières possibles. Ce travail vous sera communiqué. Vous avez raison, globalement, sur les retards dans

partenaires du logement social. Il faut avoir en tête que ce comité relève d'un décret d'application prévu par l'ordonnance du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction.

le retard partiel et une volonté de suspension sur certains sujets. Cette explication ne vaut pas spécifiquement pour le comité des partenaires du logement social, mais il est vrai que la mobilisation des services sur la préparation de la loi ÉLAN leur a fait un peu lever le pied

cette affaire est évidemment très importante -que le Gouvernement devrait nous transmettre en application de l'article 4 de la loi de programmation militaire de 2013. Nous le réclamons chaque année. Il y a trois ans, notre commission a même été obligée de se substituer Gouvernement pour évaluer les efforts consentis. Nous souhaitons vivement que le Gouvernement remplisse son obligation. Pourquoi ? Je rappelle brièvement la procédure : en application de l'article 35 de la Constitution, c'est le chef de l'État qui engage

dans votre hémicycle lors de l'examen de la LPM. Elle est prête à venir présenter le bilan annuel politique et opérationnel des OPEX, à votre convenance, dans un cadre un peu différent de celui-ci.

de santé sont essentielles pour l'évolution des prises en charge des patients, surtout dans un contexte de désertification sanitaire de plus en plus prégnante. L'application de cet article dépend évidemment de négociations qui paraissent difficiles. Pourriez-vous, monsieur le secrétaire d'État, nous indiquer l'état d'avancement de ces négociations et les principaux termes de celles-ci ? notre responsabilité est grande sur la question de l'amiante. Le repérage amiante avant travaux, pour lequel un décret a été pris, n'est toujours pas effectif, faute des arrêtés nécessaires. C'est un problème de santé publique extrêmement important. Quel est, monsieur le secrétaire d'État, l'avancement de ce dossier ?

dans un premier temps, la pratique avancée pour la profession d'infirmière, en fixant comme objectif une entrée en formation dès la prochaine rentrée universitaire. Le dispositif réglementaire est composé d'un décret en Conseil d'État et de deux arrêtés définissant le périmètre de compétence

dès septembre 2018. En ce qui concerne la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, 6 arrêtés seront nécessaires pour l'application complète du dispositif de repérage de l'amiante avant travaux, dont l'entrée en vigueur était prévue au plus tard au 1 octobre 2018. Votre alerte va dans le bon sens. Il est nécessaire que l'on puisse progresser sur ce sujet et le Gouvernement est mobilisé en ce sens. Aujourd'hui, seul l'arrêté concernant le domaine des immeubles bâtis

l'enseignement supérieur français, il faudrait préalablement qu'un décret fixe la liste des formations dans lesquelles l'admission en seconde année du deuxième cycle conduisant au master peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. Chacun ici est bien conscient des raisons pour lesquelles le Gouvernement a souhaité d'abord s'attaquer au chantier de l'orientation des étudiants, mais ne perdons surtout pas de vue la mise en oeuvre de la sélection lors de la poursuite des études. S'agissant de la loi visant à préserver l'éthique du sport, sport, plusieurs textes manquent encore pour son application. Je pense, notamment, au décret relatif au droit à l'image des sportifs. Après une période d'hésitation, voire de réticence, j'ai cru comprendre que ce texte était désormais sur les rails. Peut-être pourriez-vous nous en dire plus, monsieur le secrétaire d'État, et nous apporter des précisions ? Au-delà de ces deux textes qui ont été adoptés lors de la session 2016-2017, nous félicitons de la parution de la quasi-intégralité des mesures d'application de la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, pour laquelle le Sénat a joué un rôle important- le texte avait été voté pratiquement à l'unanimité en juillet 2016.

Je pense, par exemple, au permis de faire ouvert en matière d'urbanisme à titre expérimental, que le nouveau gouvernement a souhaité généraliser avant même la mise en place de l'expérimentation. Ce choix politique différent est, bien sûr, le signe de notre vie démocratique ... En revanche, le décret relatif au service public d'archives datant de mai 2017 laisse entière la définition du service public des archives, renvoyée bien sûr au décret lors de nos débats parlementaires. Mais nous avions souhaité, à l'époque, que soient établis

dans un trop grand nombre de situations, une méconnaissance, encore une fois, de la volonté du législateur. C'est le cas pour les emplois de docteur dans les corps de fonctionnaires de catégorie A.

de la notion de service public d'archives, le décret prévoit qu'un « service public d'archives a pour missions de collecter, de conserver, d'évaluer, d'organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur et de diffuser des archives publiques ». C'est sur cette base que nous devons travailler.

le bilan est loin d'être satisfaisant puisque, sur les 39 mesures d'application prévues, seules 13 ont été prises au 31 mars dernier, soit un taux d'application de 33 %. De plus, seulement 23 % de ces mesures avaient été prises dans les six mois suivant la promulgation. Plus grave encore, l'État a récemment été condamné, à deux reprises, par le Conseil d'État pour n'avoir pas pris certaines mesures d'application de la loi Grenelle 2, qui date de 2010. Il s'agit de mesures concernant la pollution lumineuse. Dans une décision du 28 mars, le Conseil d'État a enjoint le Gouvernement de respecter ces dispositions et de prendre dans un délai de neuf mois les arrêtés nécessaires, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour. Sur la biodiversité, dans une décision du 9 mai, le Conseil d'État a aussi ordonné au Gouvernement d'édicter dans un délai de six mois un décret fixant la liste des habitats naturels à protéger. Cette injonction est également assortie d'une astreinte de 500 euros par jour.

des dix dernières années et prévoyant des mesures d'application, 10 nécessitent encore une ou plusieurs mesures réglementaires. Enfin nous constatons, comme chaque année, que plus de la moitié des rapports demandés au Gouvernement dans des dispositions législatives n'ont pas été remis au Parlement.

Le rapport sur l'impact économique de l'interdiction des sacs plastiques devrait pouvoir être remis d'ici à la fin du deuxième semestre 2018, tout comme le rapport sur le principe de la réversibilité du stockage des déchets, qui devrait également vous être remis avant la fin de cette année. Merci,

La commission des finances constate cette année un taux de mise en application des lois promulguées de 83 %, supérieur à celui de la session précédente, qui n'était que de 76 %. Elle note également des délais en amélioration : alors que, l'an passé, moins de 30 % des mesures d'application avaient été prises dans le délai de six mois, ce taux dépasse 65 Dans l'ensemble, les textes réglementaires attendus ont été publiés et sont conformes à leur objet, ce qui est un motif de satisfaction. Cependant, nous ne pouvons bien évidemment pas nous contenter de vérifier si les décrets et arrêtés sont pris dans l'année suivant la promulgation des lois, puisque certaines dispositions législatives nécessitent une mise à jour régulière de leurs mesures d'application. Je citerai, à cet égard, deux exemples. Tout d'abord, en application de l'article

Le Gouvernement entend-il mettre à jour cette liste, comme le prévoit la loi, sans attendre qu'une nouvelle affaire conduise à des révisions en urgence ? Ensuite, l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le classement des zones tendues, qui emporte des conséquences importantes dans l'application des politiques du logement, notamment pour les dispositifs fiscaux intéressant notre commission, soit révisé au moins tous les trois ans. Or sa dernière révision date du 30 septembre 2014,

de la loi. Toutefois, alors que l'entrée en vigueur de cette disposition est désormais toute proche, des instructions fiscales semblent encore nécessaires pour préciser notamment certaines dispositions transitoires.

la présidente Valérie Létard, le Gouvernement serait bien avisé d'accepter, dans la réforme de la Constitution, que les parlementaires puissent saisir le Conseil d'État pour que celui-ci décide éventuellement d'une astreinte. Le propos que vous avez tenu à l'instant laisse bien augurer

Enfin, au-delà des décrets d'application, il y a aussi les ordonnances ... Nous avons essayé de faire comprendre au Gouvernement que son idée de banque de la démocratie était parfaitement nébuleuse. C'était un objet politique non identifié. Le Gouvernement a insisté, contre notre avis,

l'ampleur du besoin, comme le Gouvernement s'y était engagé dans le cadre des échanges qui ont eu lieu, notamment au Sénat. Après des auditions et des questionnaires adressés à des milliers de candidats, elle a conclu que le problème résidait moins dans le refus de crédits pour les candidats que dans les délais pour obtenir ces crédits et dans le manque d'information des candidats sur les démarches à accomplir pour obtenir ces prêts. Le besoin semble moins

Il est désormais d'usage que la commission des affaires européennes participe de plein droit au débat annuel sur le bilan de l'application des lois. J'en remercie le président du Sénat et la conférence des présidents. C'est important, car nos collègues sont aussi très attachés à connaître et à évaluer les suites données à leurs travaux en matière européenne. En l'espèce, que sont devenues les 18 résolutions européennes adoptées par le Sénat entre le 1 octobre 2016 et le 30 septembre 2017 ? Le rapport que j'avais présenté le 20 février dernier démontre que le Sénat est influent dans les négociations à Bruxelles. En effet,

par exemple sur le plan d'investissement pour l'Europe, sur la réforme d'EUROPOL, sur la coopération policière européenne, sur les perturbateurs endocriniens ou sur le « paquet énergie propre ». Dans plus de 25 % des cas, les positions du Sénat ont été partiellement suivies, notamment sur la phase I de l'approfondissement de l'Union économique et monétaire, la politique commerciale, la simplification du droit européen ou encore l'avenir de la politique Je me félicite de cette situation, car nos résolutions européennes ont ainsi une véritable influence sur le contenu des directives et règlements adoptés, et donc, en définitive, sur la législation française qui en résulte.

si nous nous félicitons de la très bonne coopération du secrétariat général aux affaires européennes, nous souhaitons qu'il nous transmette l'année prochaine ses fiches de suivi de façon plus régulière, et plus seulement sur demande, afin que la procédure devienne véritablement banalisée, et que notre dialogue avec le Gouvernement soit fluide et permanent. C'est une demande que nous avions déjà formulée l'an passé. Deuxièmement, nous apprécions la disponibilité de la ministre chargée des affaires européennes sur le suivi de nos résolutions. Cet exercice pourrait être approfondi par des auditions thématiques de ministres- auditions conjointes avec les commissions compétentes -, pour faire régulièrement le point sur les travaux du Conseil.

lorsque ces accords sont classifiés comme des traités simples, c'est-à-dire qu'ils ne repasseront pas devant le Parlement. Or il n'y aurait rien de plus frustrant, le mot est faible, qu'on légifère à Bruxelles sur ces sujets, dont l'incidence se fera sentir sur notre vie au quotidien.

dans le cadre de négociations avec nos partenaires européens. Dans une négociation, il y a toujours le risque que d'autres soient attentifs à nos divergences pour les utiliser contre les intérêts de la France. Ce travail en amont est donc toujours très utile. S'agissant de la transmission systématique des fiches de suivi des résolutions européennes, je sais que le SGAE veille à une diffusion dans les meilleurs délais, dès que l'accord politique est intervenu au Conseil. Je vous soutiendrai dans cette démarche et je m'en ferai le relais auprès de Mme Nathalie Pour les autres résolutions, une intervention plus précoce en amont de cet accord politique ne pourrait être que partielle et prudente, étant donné les évolutions possibles du texte jusqu'à la dernière minute des négociations. Il n'empêche que les auditions de ministres sont toujours utiles,

il sera privé de tout débat en la matière. En effet, seul le Parlement européen aura la latitude, dans un traité simple, de valider ou non la proposition d'accord de libre-échange.

la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, le nombre des articles est passé de 15, dans le projet de loi initial, à 148 dans le texte final. Autre exemple de prolifération normative : la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI siècle est passée de 54 à 115 articles, avec l'insertion de 55 articles additionnels par l'Assemblée nationale en première lecture, dont les deux tiers sur l'initiative du Gouvernement.

est celui de l'argument de la célérité des ordonnances. Il ressort du rapport d'information que le délai moyen nécessaire pour la prise d'ordonnance, en tenant compte de la procédure législative de vote de l'habilitation, est de 571 jours environ. Le délai moyen des habilitations demandées lors de la session 2016-2017 est de 344 jours environ, 309 jours en excluant les quatre habilitations pour codification, alors que le délai moyen de la procédure législative pour cette même session est de 196 jours. Le recours aux ordonnances n'entraîne donc pas une effectivité plus rapide de la norme. Que comptez-vous faire, monsieur le secrétaire d'État, pour que les ordonnances soient un outil vraiment utile et efficace ?

sait quelle est la difficulté ... Je tiens à renouveler notre engagement de maintenir à un niveau élevé le taux d'application des lois, y compris pour les dispositions introduites au cours de la navette, pour lesquelles la rédaction des mesures réglementaires n'a pu, par définition, être anticipée en amont, mais pour lesquelles nous avons la même obligation

est une exigence partagée

en réponse à la confiance que nos concitoyens nous accordent, de s'assurer que le travail législatif est bien mené jusqu'à son terme. Je remercie donc tout particulièrement Valérie Létard pour son rapport, qui illustre parfaitement la continuité du travail du législateur. Ce travail s'inscrit dans un temps contraint qui n'est pas toujours correctement perçu, car l'application des lois intervient en dehors du temps médiatique. Le bilan annuel, comme plusieurs orateurs l'ont noté, fait état d'un taux d'application des lois élevé, de l'ordre de 90 %, voire un peu plus, qui s'inscrivait, l'année de leur examen, dans un contexte préélectoral. Il est d'usage de dire, lorsque le Gouvernement utilise la procédure d'habilitation à légiférer par ordonnance, qu'il le fait pour des raisons de délais. Pour une loi d'examen comme la loi dite « Macron » de 2015, dont le champ était particulièrement étendu, l'ensemble du processus, comportant la phase législative et celle de publication des décrets, a été contenu dans un délai de douze à treize mois. Pour la loi du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, d'un périmètre volontairement plus restreint, la procédure des ordonnances a été utilisée.

ne pensez-vous pas que les efforts à accomplir en matière de gain de temps doivent aussi porter sur la publication des décrets et autres textes d'application ?

45 jours se sont écoulés pour la publication des cinq premières ordonnances et l'ensemble du dispositif a tenu dans un cadre de 101 jours. Ensuite, les décrets d'application

le recours à l'ordonnance est lié au fait que le sujet sur lequel il faut légiférer est soit d'une grande complexité, soit particulièrement épineux.

Cet arrêté a ensuite été annulé et remplacé par un arrêté identique portant application de la même loi.

mais sa réponse sera sans doute celle-là. Je connais votre argumentaire, monsieur le secrétaire d'État, vous allez nous dire qu'il fallait absolument éviter le tirage au sort à la rentrée de septembre 2018. Vous savez, comme moi, que le tirage au sort était illégal ; si telle était votre seule intention, il suffisait d'appliquer la loi !

son article 15 menace la protection du patrimoine et prévoit de transformer l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, l'ABF, en avis simple pour l'installation d'antennes relais, ainsi que pour la résorption de l'habitat insalubre dans les secteurs protégés au titre du patrimoine.

À l'Assemblée nationale, le rapporteur de la commission des affaires culturelles a bien tenté de rééquilibrer un peu le dispositif par amendement, en instaurant la possibilité de recourir à un médiateur dans le cas des recours déposés contre les avis des ABF. Mais c'est cosmétique Si le texte devait être adopté en l'état, les plans de sauvegarde et de mise en valeur ou les plans de valorisation de l'architecture et du patrimoine pourraient tout simplement être contournés, au prétexte de lutter contre l'habitat insalubre.

Sur quel bilan de la loi LCAP le Gouvernement se fonde-t-il pour remettre aujourd'hui en cause les équilibres de protection patrimoniale de ce texte ?

les missions de recherche des enseignants des établissements d'enseignement supérieur dans la création artistique, dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques. J'ai déjà eu l'occasion d'indiquer qu'après consultation interministérielle des organisations syndicales, il a été décidé que la réforme du statut des enseignants était nécessaire avant de prendre cette mesure.

ce qui nous intéresse en tant que législateur, c'est, au-delà de leur mise en oeuvre effective, l'effet de l'application des lois que nous votons dans la vie de nos concitoyens. L'article 24 de la Constitution nous confie la responsabilité d'évaluer les politiques publiques. L'exercice d'aujourd'hui relève de notre mission de contrôle, mais comment contrôler efficacement sans évaluer l'effet des textes promulgués, et inversement ? J'observe qu'en mars dernier, le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale a publié un rapport, dont je partage totalement le diagnostic en ce qui qui concerne les insuffisances de l'évaluation des politiques publiques par les parlementaires, même si je peux émettre des réserves sur les solutions proposées. Celles-ci consistent en effet à externaliser un travail que nous devrions être en mesure d'accomplir par nous-mêmes, et selon des méthodes accessibles à tous. Le 19 avril, le journal a publié une tribune signée de députés de toutes tendances, dressant le même constat. Ces députés appellent à la création d'« d'« un office d'évaluation des politiques publiques, avec en son sein une unité de chiffrage transpartisane et indépendante de l'administration et des groupes d'intérêt ». C'est en substance ce que je présentais le 7 mars dernier, en séance publique, devant notre Haute Assemblée, en proposant un conseil parlementaire d'évaluation des politiques publiques et du bien-être,

du contrôle et de l'évaluation parlementaires dans ses formes actuelles. Je sais que des réflexions sont conduites dans les deux assemblées sur ce sujet et que vous y avez contribué par votre propre proposition de loi. J'ai moi-même été entendu la semaine dernière, à l'Assemblée nationale, par la commission des finances dans le cadre du « printemps de l'évaluation », qui vise à donner davantage de substance à l'examen de la loi de règlement. Je pense que c'est essentiel. Nous passons sept semaines,

visant à mieux protéger les transports en commun contre le risque d'attentats, et à lutter contre la fraude, les incivilités et la violence au quotidien. Or, au 31 décembre 2017, date du précédent bilan de l'application des lois, 4 mesures réglementaires d'application de la loi, sur les 11 prévues par le texte, étaient manquantes. Si deux mesures ont été prises depuis cette date, deux mesures d'application prévues par l'article 18 de ladite loi étaient toujours manquantes au 31mars dernier. Je rappelle que l'application de l'article 18 doit notamment permettre le croisement des fichiers informatiques de fraudeurs avec ceux des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale. Elle est donc importante au regard de la mise en oeuvre effective de la loi. ailleurs que les demandes des exploitants et les renseignements communiqués en réponse transitent par l'intermédiaire d'une personne morale unique. Or la définition des modalités d'application de ces dispositions a été renvoyée à un décret en Conseil d'État, non pris au 31 mars dernier. Je regrette, par ailleurs, que n'ait pas été pris l'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des finances et des transports, prévu par ce même article 18, afin de déterminer le nombre maximal des agents de de la personne morale unique spécialement habilités pour accéder aux renseignements communiqués aux exploitants. J'ai attiré, en son temps, l'attention du Gouvernement sur ces retards d'application au travers d'une question écrite en date du 15 mars dernier.

tenter d'être un peu plus précis, mais j'assume le fait que cette réponse n'est pas à la hauteur de l'ambition parlementaire. Sur les quatre mesures d'application qui manquaient au 31 mars 2017, deux mesures ont depuis été prises, de sorte qu'il n'en reste plus que deux

manque actuellement deux mesures d'application de l'article 18 de la loi précitée : un décret en Conseil d'État visant à préciser les modalités selon lesquelles les exploitants des sociétés de transports publics pourront, dans le cadre d'une transaction, obtenir des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale des informations sur les contrevenants ; un arrêté visant à déterminer le nombre des agents de la personne morale unique chargés de collecter ces informations et pouvant y accéder. Ce projet de décret a fait l'objet d'une saisine du Conseil d'État le 26 janvier 2017 et a nécessité, en parallèle, une consultation de la CNIL. L'avis de cette intervenu en février 2017, donc très rapidement, après des modifications substantielles qui nécessitaient une saisine rectificative, laquelle n'a pu intervenir dans des délais raisonnables. Le Conseil d'État s'est finalement dessaisi de ce texte. C'est la raison pour laquelle la procédure doit être reprise de zéro. Votre question est une alerte, monsieur le sénateur, comme elle l'a été pour les services du ministère concerné.

La séance est reprise. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Jean-Claude Boulard, qui fut sénateur de la Sarthe de 2014 à 2017.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 L'ordre du jour appelle le débat sur le transport fluvial à la suite de la présentation du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures du 1 février 2018, organisé à la demande du groupe Les Républicains. Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur de la demande du débat dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.

on le dit, la mer semble de plus en plus être une sorte de prolongement de la terre, le fleuve est finalement une avenue, une artère, une veine irriguant tous les territoires avec une dimension éminemment européenne. S'il existe un fait maritime, il existe aussi une réalité fluviale ! À la mer, le commerce du lointain, au fleuve, l'acheminement dans les terres. Du bassin rhénan à la Provence, des Flandres à la Ligurie Mais notre vieux et beau pays, irrémédiablement centré sur sa capitale, Paris, est pourtant irrigué en toutes régions par d'importants cours d'eau. L'Europe continentale du Nord, pionnière du fluvial, se présente comme une longue plaine entre mer et montagne. Quelque part, le destin de l'Europe s'y est inscrit en favorisant les échanges par voie navigable. La géographie fluviale française se concentre autour de trois axes majeurs, commercialement stratégiques : l'axe Seine-Nord-bassin rhénan ; l'Ouest, et son grand bassin fluvial atlantique ouvert sur l'océan, connecté aux ports de la façade ; enfin, l'axe Rhône-Saône vers la Méditerranée.

Nos villes anciennes, capitales régionales, sont toutes associées aux cours d'eau. Avec l'écluse, puis les canaux de jonction, Henri IV a été le précurseur du développement économique des territoires par la navigation intérieure. Cette volonté existera pendant trois siècles avant la raréfaction des investissements et un entretien en déclin, notamment durant ces dernières décennies. Pour ce qui concerne la situation actuelle, je laisse à mes chers collègues le soin d'énumérer les chiffres clés du transport fluvial, en établissant les forces et les faiblesses de ce mode Pour ma part, je souhaite poser simplement les bases d'un débat utile parce qu'il est nécessaire de tirer le meilleur parti de nos 8 000 kilomètres de voies navigables. Ce débat doit permettre de faire émerger des propositions concrètes, des perspectives économiques et de consolider le calendrier. Nous attendons du Gouvernement qu'il nous éclaire sur les choix stratégiques qu'il souhaite opérer et qu'il nous indique s'il entend s'appuyer sur les recommandations du Conseil d'orientation des infrastructures. Un mot sur la réalité actuelle : le secteur du fret, malgré un recul quantifiable, a un besoin croissant de personnel qualifié. N'oublions pas que près de 5 000 personnes en France vivent directement du transport fluvial. Cela signifie que l'on doit mettre aussi l'accent sur la formation, à l'instar de l'apprentissage proposé par le Centre de formation d'apprentis de la navigation intérieure situé au Tremblay-sur-Mauldre, dans les Yvelines, offrant des débouchés variés aux jeunes : de matelot à commandant ou chef d'entreprise de batellerie artisanale. La prochaine loi sur la formation professionnelle

Nous attendons du Gouvernement qu'il se positionne clairement sur la question. Un euro investi dans nos voies navigables est un euro utile pour le développement de l'activité fluviale. D'autres pays l'ont compris depuis des siècles : les connexions des ports avec l'sont cruciales. La Belgique et les Pays-Bas ont prospéré bien avant le siècle d'or à partir de cette réalité fluviale, dont la République des Provinces-Unies, née de l'Union d'Utrecht signé en 1579, sut tirer un profit retentissant en se hissant au rang de première puissance commerciale au monde. Aujourd'hui encore son économie énergique y trouve sa source. Application concrète : à Utrecht, cette célèbre ville, depuis 2012, des navires électriques assurent une partie du fret et du ramassage des ordures sur un canal datant du XIIsiècle. À Amsterdam, un célèbre transporteur utilise un bateau de livraison. Comparaison ne vaut pas raison, surtout avec la France dans ce domaine au regard de géographies si différentes en matière fluviale et maritime. Pourtant, tous nos grands ports français sont aux avant-postes d'un fleuve, donc du pays de l'intérieur qu'ils irriguent depuis des temps immémoriaux. Comment répondre à la complémentarité des usages ? En donnant un nouvel élan à la logistique et au transport de marchandises sur le grand gabarit, en accroissant et en offrant une meilleure visibilité au tourisme fluvial de petit gabarit. Comment tirer le meilleur parti de l'hydraulique, notamment dans les territoires ruraux- risques, biodiversité, alimentation en eau ? Une modernisation des voies navigables Il faut investir d'urgence et mener rapidement à leur terme des projets comme la liaison Seine-Escaut, le canal Seine-Nord avec un gabarit européen. Il faut relier la Normandie et la région parisienne au Benelux grâce à une voie navigable à grand gabarit- c'est de l'aménagement du territoire. Or, aujourd'hui, les grands projets d'intérêt public sont contrariés par des minorités agissantes- pensons à Notre-Dame-des-Landes -, malgré toutes les procédures légales et démocratiquement validées. De quoi susciter quelques inquiétudes pour relancer l'aménagement du territoire, ce qui est d'intérêt public.

Quelle que soit l'inspiration qui nous anime, il s'agit non pas d'écrire un roman initiatique sur le charme fluvial, la batellerie et la traversée fantastique de la France par ses cours d'eau, mais plutôt de refonder nos pratiques et nos usages, nourris d'une volonté d'étendre le rôle commercial de nos fleuves dans une dimension européenne.

ère, bien au-delà des rimes du général de Gaulle lorsqu'il écrit en 1963 « sur ceux qui posent » : « Dans les vases clos des [ ...] débats, [ne soyons pas seulement] ceux qui exposent, [ ...] supposent, [ ...] opposent », mais plutôt « ceux qui proposent » et « transposent ». À nous d'écrire une nouvelle feuille de route en favorisant le report des marchandises vers le mode de transport fluvial, et nous aurons rendu à nos fleuves leur utilité économique en respectant leur majesté naturelle. Mais surtout, il faut lever un obstacle majeur : l'absence d'interconnexions entre nos bassins fluviaux. Voilà le véritable défi ! Après le débat, nous passerons ensuite, je l'espère, au travail. La

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de ce nouveau débat sur les travaux du Conseil d'orientation des infrastructures, le COI, au sein de la Haute Assemblée qui fait écho à nos échanges sur les lignes ferroviaires à grande vitesse, ainsi que sur la politique en matière d'infrastructures routières. Débattre du fluvial, c'est d'abord parler d'aménagement du territoire tant nos voies d'eau naturelles ou artificielles contribuent à dessiner la carte de nos territoires. Autour d'elles coexistent différentes infrastructures et usages : quais industriels, plateformes logistiques, ports de plaisance, activités nautiques, hydroélectricité, irrigation, prélèvements industriels ou promenades. Débattre du fluvial, c'est aussi souligner les enjeux environnementaux qui concernent toutes les voies d'eau, et la forte valeur patrimoniale de certains ouvrages, à commencer par l'ensemble du canal du Midi, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est donc naturellement évoquer le tourisme fluvial et la plaisance qui constituent des activités en plein essor. Débattre du fluvial, c'est enfin et surtout parler de transport de marchandises, d'un mode complémentaire à la route et au fer, d'un mode sûr, non saturé, propre : un convoi fluvial, c'est aujourd'hui 200 camions en moins sur nos routes. Toutefois, la place du fret fluvial dans notre économie n'est pas à la hauteur de ces avantages ... Loin de là ! ... puisqu'il représente moins de 3 % du transport de marchandises. Une partie de l'explication est géographique : le linéaire du réseau fluvial est bien plus faible que celui du réseau ferroviaire ou routier. Une autre tient à l'état préoccupant de notre réseau Il est clair que ce dernier est aujourd'hui vieillissant, et qu'il est nécessaire d'engager un effort important pour stopper sa dégradation et assurer sa régénération. Pour maintenir les fonctionnalités liées au transport tout en assurant la gestion hydraulique, l'investissement nécessaire pendant la prochaine décennie est bien supérieur aux montants engagés par VNF au cours des dernières années. Comme pour les réseaux routier et ferroviaire, nous devons assumer, aujourd'hui, cette situation : les investissements nécessaires ont été repoussés depuis des années. C'est ce constat qui, vous le savez, a conduit à lancer les travaux du Conseil d'orientation des infrastructures, présidé par Philippe Duron. Le rapport qui m'a été remis le 1 février dernier est le fruit d'un travail considérable. Issu d'un large consensus, il a été adopté à l'unanimité des seize membres, experts et élus, dont vos collègues Hervé Maurey, Gérard Cornu et Michel Dagbert, que je veux une nouvelle fois remercier de leur engagement. Ce travail pose les bases d'une programmation sincère, ambitieuse et réaliste des infrastructures qui sera déclinée dans le projet de loi d'orientation sur les mobilités que je défendrai prochainement devant la Haute Assemblée.

afin d'atteindre progressivement les montants nécessaires pour la remise à niveau du réseau, en tenant compte des moyens propres de VNF et des efforts que doit faire cet établissement. d'un investissement important en termes de modernisation dans les cinq ou dix prochaines années selon le scénario, pour accompagner la fiabilisation des équipements de navigation et la modernisation des méthodes d'exploitation. enfin, d'un soutien aux trois grands projets fluviaux étudiés par le COI : l'aménagement de la Lys mitoyenne, la mise à grand gabarit de l'Oise entre Creil et Compiègne et la mise à grand gabarit de la Seine amont entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine. Il est également un projet sur lequel vous êtes- je le sais -nombreux à être attentifs : le canal Seine-Nord. Je n'y insisterai pas maintenant, car je ne doute pas qu'il sera au coeur de nombreuses questions qui me seront posées. La programmation des infrastructures de transport que je présenterai au Parlement tiendra bien évidemment compte de ces orientations. La robustesse et la fiabilité des infrastructures sont en effet un préalable au développement du trafic fluvial. Une situation comme celle de la Seine amont, où les bateliers, les chargeurs céréaliers ou du BTP ont connu d'importantes restrictions de navigation ces derniers mois à la suite des dégâts occasionnés par les crues, n'est pas acceptable. Au-delà de cet objectif, d'autres efforts doivent être faits. Je pense d'abord au renforcement de la connexion entre les points maritimes d'import et d'export que sont nos grands ports et les ports intérieurs pour constituer de véritables logiques d'axes logistiques et portuaires le long des axes fluviaux. Les missions confiées par le Premier ministre au préfet Philizot sur l'axe Seine, au préfet Lalande sur l'axe Nord et à Jean-Christophe Baudouin sur l'axe Méditerranée-Rhône-Saône répondent à cet objectif. Il s'agit également d'accompagner le transport fluvial de marchandises et de passagers pour qu'il saisisse toutes les opportunités de développement économique, en surmontant quatre grands défis.

À ce titre, je me réjouis de la validation par la Commission européenne, la semaine dernière, du nouveau plan d'aide au report modal, le PARM, doté d'une enveloppe de 20 millions d'euros sur la période 2018-2022 et mis en place par VNF pour favoriser le report modal vers la voie d'eau, au travers d'une aide aux chargeurs. Le deuxième défi est celui de la transition numérique ; l'objectif est que le transport fluvial se saisisse de toutes les opportunités offertes par la digitalisation des chaînes logistiques et par la dématérialisation des procédures administratives. Le troisième défi est celui de la performance environnementale ; il convient de saisir toutes les capacités d'innovation pour que le transport fluvial se positionne comme un mode de transport propre. Le verdissement de la flotte fluviale est ainsi l'un des principaux objectifs du nouveau plan d'aides à la modernisation et à l'innovation, le PAMI, doté de 16,5 millions d'euros sur la période 2018-2022, également géré par VNF et approuvé par la Commission européenne en même temps que le PARM. Enfin, le quatrième défi est le défi social ; il s'agit d'offrir des conditions attractives d'emploi. Pour relever ces défis, le secteur fluvial français doit impérativement se rassembler, afin de mener des actions collectives impliquant les différents intervenants de la chaîne de transport. C'est pourquoi j'ai demandé au préfet François Philizot d'organiser la préfiguration d'une interprofession fluviale, avec l'ensemble des parties prenantes intéressées, la réunion de lancement aura lieu demain. Vous le voyez, nous allons conduire dans les prochaines années une politique volontaire et exigeante en faveur du mode fluvial. En cohérence avec la démarche de programmation des infrastructures et d'élaboration d'une loi d'orientation sur les mobilités que nous menons actuellement, nous avons engagé avec VNF des discussions sur le modèle économique, les ressources et les objectifs pluriannuels de cet établissement, afin d'améliorer la qualité de service et la disponibilité du réseau, d'optimiser son organisation et de maîtriser les risques. Ces démarches conduiront à un contrat d'objectifs et de performance avec l'établissement, dans lequel je souhaite que l'État s'engage sur des moyens, et VNF sur des résultats. Programmation des infrastructures de transport, projet de loi d'orientation sur les mobilités, contrat d'objectifs et de performance : voilà l'ensemble des dispositifs qui nous permettront d'établir une vision stratégique claire, avec des objectifs réalistes et sincères, afin de permettre au secteur fluvial de réussir sa transformation et son développement au service de l'aménagement du territoire et de la transition écologique. Je rappelle transition écologique. Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes maximum pour présenter sa question, suivie d'une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

Pour moi, élue de Seine-Maritime, département où Le Havre s'impose comme l'un des plus grands ports de France et d'Europe, ce sujet est prépondérant sur le plan de l'intérêt économique et environnemental de la région et du territoire national. Ce port, qui affiche un réel déficit du point de vue du transport fluvial, subit un retard important au regard des autres grands ports européens, dont Rotterdam et Anvers. En effet, la part du fluvial dans le trafic de conteneurs depuis et vers le port du Havre ne représente que 9 %, contre respectivement

de gaz à effet de serre. Ce retard tient essentiellement au manque d'infrastructures. En effet, Port 2000 a été construit sans qu'aucun accès fluvial au nouveau bassin ait été réalisé. Trois projets ont été proposés, dont celui de la construction d'une « chatière

Oui, le port du Havre a des atouts indéniables, que nous nous devons de renforcer et de développer, afin d'en améliorer la compétitivité, d'autant plus que les porte-conteneurs, de plus en plus gros, n'accéderont plus aux ports de Bordeaux ou de Nantes et transiteront par Le Havre. Lors des dernières assises de l'économie de la mer, le Premier ministre faisait mention d'une indispensable stratégie portuaire nationale pour les trois grands ports du pays, dont Le Havre. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est aujourd'hui ? La parole est à Mme la ministre.

Ce port a saisi la Commission nationale du débat public, qui a recommandé, en juillet 2017, de mener une concertation et qui a désigné une garante. Cette concertation a été lancée le 20 octobre 2017 et s'est conclue le 19 janvier Trois options ont été présentées à la concertation : la réalisation d'un accès direct en zone protégée accessible à tout type de bateau- la fameuse chatière -, l'extension du terminal multimodal et l'optimisation des solutions en place. À la faveur de la concertation, la notion de complémentarité des options a émergé. La garante a rendu son rapport le 18 février dernier. Grâce à cette concertation, le maître d'ouvrage, le grand port maritime du Havre, a adopté lors de son conseil de surveillance de mars dernier un plan de développement du fluvial autour de cinq grandes priorités. Par ailleurs, il a intégré le projet de chatière dans le programme d'investissement en cours d'élaboration. Des discussions se déroulent actuellement sur la priorisation de ce programme et feront l'objet de débats lors du prochain conseil de surveillance, qui tout état de cause, je vous confirme ma détermination à renforcer la part du transport fluvial et ferroviaire dans la desserte de nos ports. Vous l'avez souligné, étant donné le développement de porte-conteneurs de plus en plus importants, si l'on ne veut pas voir nos routes

Cette recommandation, si elle était suivie, aurait des conséquences dramatiques pour une large portion du territoire. La fermeture de ces canaux, c'est l'isolement de nombreux villes et villages qui drainent aujourd'hui des flux par le transport fluvial c'est encore l'appauvrissement de nombreux sites touristiques, privés de leurs visiteurs et délaissés par les voies de transport ; c'est enfin une perte nette de ressources pour des territoires et la porte ouverte à un exode des populations. Supprimer des voies navigables, madame la ministre, c'est affaiblir notre maillage territorial. À l'heure où les débats sur la réforme ferroviaire se concluent, vous avez saisi toute l'importance du maintien d'un aménagement durable de notre territoire, en souscrivant à la préservation de dessertes isolées ou rurales. En 2016, la France ne représentait que 6 % du trafic fluvial européen, alors que près de 20 % du linéaire des voies européennes se situent dans les limites de l'Hexagone. Cela marche en Cela marche en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne ; pourquoi pas en France ? Ne renonçons pas à la mise en oeuvre du canal Seine-Nord et à la préservation des petits canaux.

au contraire, de développer le réseau de transit fluvial international et de longue distance, pour encourager nos entreprises de transport à plus de compétitivité et à une plus grande intermodalité. La parole est à Mme la ministre.

dont l'objectif serait de fermer à la navigation les 20 % du réseau les moins circulés, afin de concentrer les dépenses sur la sauvegarde du patrimoine le plus emprunté Il est vrai que certaines voies navigables, en raison de leur gabarit ou de leur nombre important d'écluses, ne sont plus adaptées au transport de fret et n'ont pas non plus de potentiel touristique. Ces voies sont donc très peu ou non circulées. Dès lors, le projet stratégique de VNF, adopté en 2015 après concertation, a prévu, pour certaines voies, une offre de services saisonnalisée ou une ouverture uniquement sur demande.

Ce serait une approche erronée de penser que la dénavigation permettrait de réduire les investissements, puisque, aujourd'hui, nous n'atteignons pas ce rythme d'investissement de 245 millions d'euros par an. En tout état de cause, l'option consistant à fermer 20 % du réseau sans aucune autre forme d'analyse que celle de la fréquentation n'est pas envisageable ni envisagée. Pour autant, la fermeture de certains tronçons peut être considérée, mais elle devra nécessairement être précédée d'une réflexion sur la cohérence du maillage du réseau, sur le potentiel industriel et touristique et sur les projets des collectivités locales. Je veux, à ce titre, citer un exemple, en saluant le projet de réouverture du canal de la Sambre à l'Oise,

pourquoi est-il à la peine ? Pour des raisons économiques et structurelles, tout d'abord : le transport fluvial est encore insuffisamment rentable du fait de la vétusté de certaines parties du réseau et de défauts d'interconnexion, en son sein ou avec les autres modes de transport.

140 millions d'euros à l'échelle nationale, soit l'équivalent du budget d'investissement du seul département du Pas-de-Calais ... Pour des raisons liées à la faiblesse du portage politique, ensuite ; avec des renoncements, tel celui du canal Rhin-Rhône, avec l'adoption de mesures favorables au transport routier,

Le niveau d'investissement de VNF s'est réduit, passant de 157 millions d'euros en 2013 à 138 millions d'euros en 2018. Ce montant d'investissement est très en deçà du niveau nécessaire à la seule régénération du réseau fluvial, estimé à 245 millions d'euros par an, hors modernisation et développement. Vous le savez, le réseau fluvial est vieillissant et fragile, comme en témoignent les épisodes de crues de 2016- je pense à la rupture d'une digue sur le Loing, affluent de la Seine -et de 2018- d'importantes interruptions de navigation ont

en dix ans, pour financer le socle d'investissement de régénération du réseau, mais aussi un montant de 330 millions d'euros sur cinq ans pour la modernisation des méthodes d'exploitation, nécessaire à la fiabilisation du réseau à grand gabarit et aux gains d'exploitation de productivité de l'établissement. Pour ce faire, le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures envisage la transformation de la taxe hydraulique en une redevance domaniale, afin de sécuriser juridiquement le dispositif et de conforter la ressource financière, ainsi que la dynamisation des recettes propres de l'établissement et les efforts de productivité pour réduire les dépenses. Ces orientations trouveront naturellement leur place dans le projet de loi d'orientation sur les mobilités, notamment dans son volet programmation. Par ailleurs, je l'ai indiqué, un contrat d'objectifs et de performance permettra de définir une trajectoire claire, réaliste et sincère pour l'établissement public pour les prochaines années. La parole

dont 1 600 kilomètres pour les grands gabarits, la France semble disposer des atouts nécessaires au développement du transport fluvial. Malheureusement, les routes fluviales restent sous-exploitées. Au Havre, ville dont je suis et dont ma collègue Nelly Tocqueville vient de parler, il est clair que le report sur les voies fluviales reste extrêmement faible, puisque seuls 9 % des conteneurs sont acheminés par la Seine.

dit, la qualité des infrastructures n'est pas la seule faiblesse du transport fluvial. Le coût du transport combiné constitue aujourd'hui son premier frein. en France, contrairement aux ports du nord de l'Europe, les opérateurs de transport fluvial doivent supporter seuls le coût des ruptures de charge, ce qui alourdit la facture du transport de marchandises

concurrentiel. Madame la ministre, comment garantir un écosystème attractif qui permette au transport fluvial d'avoir toute sa place dans le transport combiné des marchandises en France, à l'instar de ce qui existe dans les ports du nord de l'Europe ? est à Mme la ministre. Madame la sénatrice, la compétitivité du transport fluvial est effectivement essentielle si nous voulons favoriser le report modal pour le transport de marchandises. Le transport fluvial est naturellement affecté par les surcoûts liés aux acheminements terminaux, dans la mesure où l'infrastructure fluviale n'est pas présente sur l'ensemble du territoire. La maîtrise du foncier en bord à voie d'eau est un élément clef pour permettre un report modal de la route vers la voie d'eau. Afin de disposer de leviers supplémentaires pour réserver les terrains en bord de voie d'eau nécessaires à l'activité fluviale, on envisage d'insérer dans le projet de loi d'orientation sur les mobilités des mesures visant à donner la possibilité à VNF de se voir déléguer le droit de préemption urbain des communes. Dans les zones où les besoins fluviaux sont avérés, cette mesure permettrait à VNF de travailler avec les conseils municipaux sur les enjeux de la voie d'eau, de sensibiliser ces assemblées à son utilisation et de créer une dynamique très positive au plus près des territoires. Par ailleurs, deux dispositifs d'aides sont prévus pour encourager le report modal sur la voie d'eau. Le premier est le plan d'aide au report modal, doté, je le disais, de 20 millions d'euros pour la période 2018-2020 ; il doit permettre d'accompagner de nouveaux trafics, jugés stratégiques, jusqu'à leur phase de maturité. Il se traduit par une aide aux chargeurs selon trois modalités : réalisation d'études préalables, expérimentation et acquisition d'équipements, qu'il s'agisse d'infrastructures ou d'outillage. En complément, le second dispositif est l'aide au surcoût de transbordement pour le transport de conteneurs par voie ferroviaire et fluviale, le dispositif d'aide à la pince que vous évoquiez. Très prochainement, je pourrai présenter le nouveau dispositif qui s'appliquera aussi bien au ferroviaire qu'au fluvial. Des annonces seront faites rapidement à ce sujet.

ont jusqu'à présent toutes échoué. Les infrastructures ferroviaires et fluviales sont loin d'être utilisées à la hauteur de leurs capacités en matière de fret, et ce malgré les nombreux avantages qu'elles présentent. La France doit se doter d'infrastructures et de services de fret performants, et identifier le mode de transport le plus pertinent pour acheminer les marchandises, que ce soit par la route, par le réseau ferré ou par les voies navigables. Cela doit se faire sur la base d'une vision globale des capacités et des opportunités, afin de ne pas superposer frets ferroviaire et maritime. Face à ce constat, les conclusions du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures invitent à réinventer les dynamiques de logistique et à développer le fret ferroviaire et fluvial. domaine du transport fluvial, il faut lutter contre le vieillissement du patrimoine, développer et moderniser les équipements des ports fluviaux à enjeux, et inciter les acteurs à utiliser ce mode de transport de marchandises.

ces ports bénéficient aujourd'hui des retombées des constructions d'infrastructures et de logement du Grand Paris. De son côté, le port du Havre a présenté, voilà deux mois, un plan d'investissement de plusieurs centaines de millions d'euros,

de plus en plus grands, des mesures concrètes et ambitieuses sont nécessaires. Quelles seront vos propositions pour une modernisation réelle et efficace de l'axe Seine ? La parole est à Mme la ministre. est à Mme la ministre. Monsieur le sénateur, le bassin de la Seine constitue effectivement l'axe majeur du trafic de fret fluvial en France, concentrant plus de 50 % du trafic français. Vous l'avez souligné, cet axe relie les grands ports du Havre, de Rouen et de Paris.

VNF mène actuellement un important programme de régénération et de modernisation des ouvrages, prévu jusqu'en 2027, qui représente plus de 250 millions d'euros d'investissement. Il s'agit de sécuriser, de fiabiliser mais aussi, pour certains ouvrages, d'augmenter le gabarit. Parmi ces opérations, celle de Méricourt est la plus emblématique : la moitié du trafic circulant sur le bassin de la Seine passe par les écluses de cette ville qui accueillent plus de 250 bateaux par semaine. Or le vieillissement de ces écluses, dont j'ai pu me rendre compte sur place, impose une reconstruction quasi intégrale, tout en maintenant la navigation pendant toute la durée des travaux. Pour cette opération, cofinancée par la région d'Île-de-France au titre des contrats de plan État-régions et par l'Union européenne, la phase de dialogue compétitif est en cours, pour un marché de conception-réalisation. En complément, compte tenu des fragilités révélées ces derniers mois partie Seine amont, VNF élabore un plan d'investissement pluriannuel d'urgence sur ce secteur, de manière à renforcer la robustesse de l'itinéraire. Les conclusions de la mission de M. Philizot pour la modernisation de la gouvernance portuaire de l'axe Seine seront également présentées prochainement.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous connaissons depuis de nombreuses années une situation dans laquelle les voyants de tous les secteurs des transports sont au rouge, avec une augmentation des émissions de gaz à effet de serre due à la progression de tous les trafics routiers au détriment du ferroviaire et du fluvial. Pourtant, vous en conviendrez, pouvoir naviguer sur des milliers de kilomètres, c'est la richesse de la France. Avec 8 500 kilomètres de voies navigables, ce réseau fluvial est le plus long de l'Europe. Alors qu'il est un atout, notre réseau demeure mal exploité, quand il n'est pas totalement inexploité. Cette situation, due aux politiques du tout routier, conduit, d'une part, à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, et, d'autre part, à une saturation de nos routes- il n'y a qu'à faire un trajet

Dans le département de la Loire, la ville de Roanne et le canal Roanne-Digoin ont tous les atouts pour contribuer au développement du fluvial : la chambre de la batellerie est prête à affréter des produits, des industriels roannais sont intéressés, la majorité des élus locaux ont émis un avis favorable, les vignerons de la Côte-roannaise sont prêts à véhiculer leur vin par péniche et Voies navigables de France a réalisé d'importants travaux sur le canal

Il fait donc vraiment partie des travaux du Conseil d'orientation des infrastructures de programmer des moyens suffisants pour la régénération et la modernisation de nos itinéraires fluviaux. Peut-être faudra-t-il avoir une politique centrée aussi sur les quelques itinéraires les plus prometteurs du point de vue du fret fluvial- c'est le sens des questions posées dans le rapport sur l'éventuelle fermeture au trafic de certaines voies

de notre réseau fluvial. Je mentionnais l'axe Seine ; on a aujourd'hui à portée de main une autoroute fluviale, si je puis dire, qui ne demande qu'à être modernisée pour permettre un report important de la route sur le fleuve. d'autres canaux sont de plus petite importance. Vous mentionnez en particulier le canal de Roanne à Digoin- un canal latéral à la Loire datant du XIX siècle.

En revanche, cet axe connaît une dynamique touristique certaine, et je pense que le département de la Loire est très mobilisé pour y favoriser le développement du tourisme fluvial. Les

D'un point de vue environnemental, les solutions les plus vertueuses sont donc aussi les moins exploitées. Quand on sait que les volumes des échanges sont en constante augmentation, il convient d'orienter les investissements en accord avec nos objectifs environnementaux. Nous avons déjà eu l'occasion de débattre des problématiques du fret ferroviaire. Pour ce qui est du fret fluvial, ce même rapport, faisant référence à l'audit réalisé par MENSIA Conseil, évalue le volume d'investissement pour remettre en état le réseau fluvial à hauteur de 245 millions d'euros en moyenne par an sur une période de dix ans.

Mes questions sont simples : pour être en parfaite adéquation avec l'accord de Paris, avez-vous inclus ce report modal vertueux dans votre stratégie ?

est à Mme la ministre. Madame la sénatrice, en 2017, un peu plus de 52 millions de tonnes de marchandises ont été transportées par voie d'eau, ce qui représente 6 700 millions de tonnes-kilomètres. Si ce volume avait été acheminé par la route, cela aurait représenté 470 000 tonnes de CO2, alors que le transport fluvial émet en moyenne trois fois moins de dioxyde de carbone que le transport routier. Par conséquent, favoriser le report modal vers la voie d'eau permet intrinsèquement de réduire ces émissions, donc de contribuer à la réalisation des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans l'accord de Paris. Je partage tout à fait votre avis : il faut aller plus loin. Pour se positionner comme un mode de transport plus propre et une solution crédible à la congestion routière, le fret fluvial doit offrir des solutions logistiques performantes. Cela passe d'abord par la régénération de notre infrastructure fluviale et sa modernisation. Comme je l'ai évoqué, le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, s'appuyant sur l'audit qui a été mené, évalue à une centaine de millions d'euros de plus par an les besoins liés à la régénération et, par ailleurs, à

cette transition, plusieurs dispositifs d'aide sont prévus. Premièrement, le PAMI, le plan d'aides à la modernisation et à l'innovation, permet d'accompagner la transition énergétique de la flotte fluviale de marchandises.

Je me réjouis que vous y fassiez régulièrement référence, tant le travail réalisé par celui-ci a été d'une grande ampleur, même s'il n'a pas été exhaustif. En effet, je dois le reconnaître,

Les études prospectives réalisées par Voies navigables de France démontrent la possibilité de quadrupler l'ampleur du trafic fluvial sur cet axe, pour passer à 15 millions de tonnes de marchandises transportées par an à l'horizon 2020.

à respecter les obligations fixées par l'Union européenne. De même, ils souhaitent avoir toutes les garanties d'une présence pérenne des représentants de l'État dans la gouvernance de la société de projet. Monsieur le sénateur, je peux vous l'assurer, nous travaillons avec les élus locaux sur ce projet, qui est effectivement un projet d'ampleur, d'ampleur, par son montant- 4,9 milliards d'euros -, mais aussi parce qu'il doit assurer la connexion du bassin de la Seine au réseau des voies navigables du nord de l'Europe pour les convois fluviaux à grand gabarit. Vous le savez, le Premier ministre a fixé, en octobre dernier, les orientations permettant la poursuite de ce projet. Il s'agit notamment de faire évoluer la gouvernance de la société de projet vers un établissement public local permettant de transférer le pilotage financier et opérationnel, ainsi que la maîtrise des risques du projet aux collectivités territoriales. Pour sa part, l'État a confirmé son engagement à hauteur de 1 milliard d'euros, un emprunt de long terme de la société de projet, dont les annuités pourraient être financées par des taxes nationales à assiette locale affectées à la société de projet. Les travaux autour de la régionalisation de la société de projet, laquelle nécessite des dispositions législatives qui seront proposées dans le projet de loi d'orientation sur les mobilités, sont en voie de conclusion. L'objectif est que cette régionalisation soit effective dans le courant de l'année 2019, comme j'ai pu le confirmer récemment à M. Xavier Bertrand. Parallèlement, les échanges avec les collectivités territoriales se poursuivent pour consolider le plan de financement, sur la base des orientations fixées par le Premier ministre. La parole est à M. Didier

Cette différence s'explique, en partie, par le manque d'investissement dans le réseau fluvial et par l'absence de développement d'une vraie politique de transport de marchandises intermodale. En 2009, un audit généralisé du réseau a permis d'évaluer l'état fonctionnel de la quasi-intégralité des ouvrages et d'en déduire les besoins d'investissement pour le garder tel qu'il Pourtant les investissements n'ont cessé de diminuer. En cinq ans, VNF a perdu un quart de ses ressources d'investissement : son budget est passé de 200 millions d'euros à 130 millions d'euros en 2017, alors qu'un audit récent a évalué l'investissement nécessaire

vous avez apporté tout à l'heure des éléments de réponse à cette question légitime des moyens à mettre en oeuvre. C'est une avancée, mais c'est encore et toujours insuffisant. Les hésitations du Président de la République sur le projet de canal Seine-Nord montrent à quel point le transport fluvial n'apparaît pas aujourd'hui comme une priorité. À l'heure où les questions de lutte contre le réchauffement climatique et la pollution sont déterminantes, à l'heure où les routes sont saturées et où les temps d'acheminement des marchandises augmentent, à l'heure où nos voisins européens misent sur le multimodal,

Je pense à la rupture de digue sur le Loing en 2016 ou aux blocages récents des installations de la Seine amont. Effectivement, l'audit réalisé sur l'état de nos infrastructures fluviales a permis de conclure qu'il faudrait 245 millions d'euros par an pendant dix ans pour régénérer le réseau fluvial, après des décennies de sous-investissement. Vous me demandez pourquoi nous n'investissons pas massivement dans le transport fluvial.

de loi de programmation des infrastructures que j'aurai l'occasion de vous présenter prochainement. Je pense que nous devons, en effet, être en mesure de proposer un scénario de rattrapage de l'état de nos infrastructures, qu'elles soient ferroviaires- nous les avons évoquées dernière -, routières ou fluviales. S'agissant des infrastructures fluviales, effectivement, le montant que VNF a consacré à la régénération ces dernières années n'est pas du tout à la hauteur des besoins qui ont été identifiés. Il manque quelque 100 millions d'euros par an pour assurer le maintien en état de notre patrimoine, sans compter les sommes nécessaires pour le moderniser. Vous le voyez, nous aurons des choix

Pourtant, ce mode de transport devrait être fortement développé à l'avenir, tant il présente d'avantages. En particulier, il émet relativement peu de gaz à effet de serre et son développement permettrait de décongestionner un réseau routier trop souvent saturé. Toutefois, il n'y aura pas de report modal significatif vers le transport de marchandises sans une volonté politique forte et une stratégie cohérente. Les chantiers sont nombreux relance des investissements dans un réseau vieillissant, développement des synergies avec les ports ... Telles sont les conclusions du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures. L'État a d'ores et déjà pris des mesures en ce sens, ce dont on ne peut que se réjouir.

Or actuellement les entrepreneurs souhaitant faire transporter leurs marchandises sont insuffisamment informés sur l'offre existante en matière de transport fluvial, ainsi que sur les avantages propres à celui-ci sa fiabilité, sa sécurité, le réseau de voies navigables de plus de 6 700 kilomètres qui parcourt notre pays, sans oublier, bien sûr, les avantages sur le plan écologique. Le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures dévoilé le 1 février dernier dresse ce constat, en évoquant, parmi les propositions en faveur du développement du transport fluvial, l'incitation des chargeurs et des transitaires à prendre en compte ce mode de transport, par des modes de communication adaptés ». Le Gouvernement partage-t-il cet avis et, si oui, quelles mesures compte-t-il prendre en ce sens ? La parole est à Mme la ministre. est à Mme la ministre. Monsieur le sénateur, effectivement, le transport fluvial est aujourd'hui encore trop peu connu des donneurs d'ordre du transport de marchandises, aussi bien des chargeurs, des logisticiens que des acteurs publics. De nombreuses actions ont été engagées, en particulier par VNF, pour améliorer la visibilité et la prise en compte de la voie d'eau par les donneurs d'ordre. S'agissant des chargeurs et des logisticiens, la connaissance du transport fluvial passe d'abord par la formation des acteurs à ce mode de transport. À ce titre, VNF intervient dans une vingtaine de formations liées à la logistique et au transport et a noué, depuis 2011, un partenariat avec le Groupe Sup de Co La Rochelle,

permet d'accompagner de nouveaux trafics par voie d'eau, jugés stratégiques, jusqu'à leur phase de maturité. Il se traduit par une aide qui intervient selon trois modalités : réalisation d'études préalables, expérimentation ou acquisition d'équipements. toutes ces actions devraient pouvoir être assumées, de manière collective, par la profession du transport fluvial. C'est pourquoi j'ai demandé au préfet François Philizot de préfigurer une interprofession fluviale avec l'ensemble des parties prenantes intéressées.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans son rapport, le Conseil d'orientation des infrastructures a étudié l'opportunité de la construction d'infrastructures fluviales nouvelles pour notre pays, à l'exception du canal Seine-Nord, qu'il a écarté de son champ d'analyse, considérant que ce dernier était déjà acté par ailleurs. Je me réjouis de cette déclaration, qui confirme la réalisation du canal, projet essentiel pour notre pays et pour le développement du transport fluvial. C'est par ailleurs un élément central de la liaison fluviale européenne Seine-Escaut, classée comme prioritaire par le réseau transeuropéen de transport, même si de nombreuses interrogations subsistent quant au positionnement du Gouvernement, en particulier sur la question du financement. Le rapport s'intéresse néanmoins à deux autres ouvrages en lien étroit avec celui du canal, pour lesquels il recommande, quel que soit le scénario envisagé, de prévoir l'engagement des travaux. d'une part, du projet MAGEO, relatif à la mise au gabarit européen de la rivière de l'Oise entre Compiègne et Creil, qui permettra ainsi la continuité de circulation des convois entre la Seine et le futur canal. La réalisation de cet aménagement est donc incontournable. Il s'agit, d'autre part, du recalibrage de la Lys mitoyenne entre Deûlémont et Halluin, à la frontière belge. Je me félicite de ces propositions. Cependant, le rapport précité ne formule que des préconisations, que le Gouvernement n'est en rien contraint de suivre- l'exemple du rapport Borloo nous l'a prouvé. Or, en l'espèce, nous connaissons les réticences du Premier ministre. Aussi, madame la ministre, considérant l'importance de ces deux projets et compte tenu des nombreux engagements et investissements déjà réalisés, pourriez-vous nous indiquer si le Gouvernement entend suivre les recommandations de ce rapport et engager les financements nécessaires à la réalisation de ces infrastructures ? La parole

de l'Oise entre Creil et Compiègne, ou projet MAGEO, d'un coût de 288 millions d'euros, constitue le débouché sud du projet de canal Seine-Nord. Elle est donc indispensable à son plein effet. Le Conseil d'orientation des infrastructures a rappelé son caractère incontournable et la nécessité de la financer, quel que soit le scénario retenu. L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique doit se dérouler à la fin de cette année. Le Conseil préconise, dans tous les scénarios, la réalisation des travaux principaux à partir de 2023.

l'aménagement de la Lys participe à la réalisation du canal Seine-Nord Europe et à la constitution du futur réseau fluvial à grand gabarit Seine-Escaut. Ce projet se situe à la fois en France, en Wallonie et en Flandre. La maîtrise d'ouvrage et les coûts ont donc été répartis entre les trois territoires. Le projet a été examiné par le Conseil d'orientation des infrastructures, qui préconise qui préconise la réalisation des travaux sur la période 2018-2022, quel que soit le scénario retenu. La participation de l'État s'élèverait à 12 millions d'euros. L'enquête publique est prévue à la fin de cette année, pour un arrêté de déclaration d'utilité publique qui sera pris au début de l'année prochaine.

Le Président de la République a souhaité rassurer sur sa réalisation d'ici à huit ans. Qu'en est-il de son financement ? Le projet est estimé à 4,5 milliards d'euros par les pouvoirs publics. L'Union européenne investira 2 milliards d'euros. Les collectivités territoriales participeront à hauteur de plus de 1 milliard d'euros. Les régions Hauts-de-France et d'Île-de-France s'engagent à une participation supérieure à 500 millions La contribution de l'État, à 1 milliard d'euros, reste encore à préciser. La participation de la région d'Île-de-France traduit une volonté de construire le Grand Paris fluvial, maillon français indispensable du projet de liaison fluviale européenne Une accessibilité la région d'Île-de-France permettrait de rejoindre les grands ports maritimes. En sortant du statut de cul-de-sac fluvial, la région d'Île-de-France deviendrait, d'ici à 2024, une autoroute pour péniches de grand gabarit, notamment entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, à même d'assurer les capacités exportatrices de la filière agricole française. Le partenariat interrégional et multimodal avec les Hauts-de-France permet d'espérer 10 000 emplois directs et indirects, une accessibilité directe pour l'importation et l'exportation de produits alimentaires et non alimentaires, une traçabilité et une sécurité accrues du fret et, surtout, une baisse du coût du transport et de la pollution. Madame la ministre, ce canal est indispensable pour que notre pays reste compétitif dans le cadre de la mondialisation des échanges. Pouvez-vous nous préciser le plan de financement sur lequel l'État compte s'engager et le calendrier retenu ? Le projet du canal Seine-Nord a besoin d'un signal fort, de l'expression d'une volonté renouvelée et d'une clarification. la ministre. Monsieur le sénateur, je vous confirme les orientations qui ont été fixées par le Premier ministre en octobre dernier s'agissant du financement du canal Seine-Nord, projet estimé à 4,9 milliards d'euros. Il s'agit de faire évoluer la gouvernance vers un établissement public local permettant de transférer le pilotage financier et opérationnel ainsi que la maîtrise des risques du projet aux collectivités territoriales. Cependant, l'État a confirmé son engagement à hauteur de 1 milliard d'euros, un emprunt de long terme de la société de projet, dont les annuités pourraient être financées par des taxes nationales à assiette locale affectées à la société de projet. Les travaux autour de la régionalisation avancent avec les collectivités concernées.

sa réalisation, quels que soient les scénarios retenus sur la période 2028-2032. Les études préalables à l'enquête publique sont en cours, dans la perspective d'une enquête publique qui pourra se tenir à l'horizon 2019. Vous le voyez, nous sommes en train de travailler sur l'ensemble de ces aménagements.

est à Mme la ministre. Monsieur le sénateur, la question de la place du transport fluvial dans notre transport de marchandises est effectivement un sujet important. Je ne peux pas me satisfaire de la place que le transport fluvial-

de formation et de sensibilisation à l'intérêt de ce mode de transport fluvial. Enfin, il faut être capable d'attirer de nouveaux chargeurs vers la voie d'eau. C'est tout le sens des dispositifs de soutien au transport fluvial, qu'il s'agisse du plan d'aides à la modernisation et à l'innovation, pour avoir, demain, un transport fluvial

Madame la ministre, je souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur la liaison fluviale à grand gabarit entre la Moselle et la Saône,

liaison Rhin-Rhône par la Moselle et la Saône dépasse le fait de relier les bassins par des canaux à grand gabarit. Il s'agit aussi d'adapter les voies aux dimensions des bateaux et de désengorger les canaux existants.

! Des études ont été entamées par l'État, nous le savons, mais, à notre connaissance, elles n'ont pas été achevées. Il est fondamental de relier la mer du Nord à la Méditerranée. J'aimerais, en conséquence, savoir, madame la ministre, où en sont les études et les discussions sur ce projet. Le Gouvernement soutient-il toujours cette mise en oeuvre ? Et si oui, quels moyens compte-t-il investir ?

Le linéaire concerné représente environ 350 kilomètres, pour un coût de l'ordre de 15 milliards d'euros. L'enjeu est de relier aux principaux réseaux fluviaux et maritimes européens les ports maritimes et le réseau fluvial à grand gabarit de l'est de la France. la France. Le coût de cette infrastructure apparaît hors de portée des financements actuellement envisageables. J'ai mentionné les besoins complémentaires et les sommes supplémentaires qu'il nous faudrait consacrer à la régénération et à la modernisation de notre réseau fluvial, sans parler des projets d'aménagement autour du canal Seine-Nord et du canal Seine-Nord lui-même et des autres besoins afférents aux projets ferroviaires ou routiers. À regarder le

Dans ces conditions, la perspective d'un débat public, initialement envisagé et qui avait fait l'objet d'une préparation entre VNF et les collectivités locales concernées, a été abandonnée

Je le rappelle, il contribuera à développer une mobilité durable dans notre pays et il est au centre de toutes nos attentions. Toutefois, vous le savez, des interrogations sur son financement persistent. Les inquiétudes portent notamment sur l'origine de la part du financement de l'État qui reste, quant à elle, à définir, même si, madame la ministre, vous nous avez donné plusieurs pistes, sur lesquelles je reviens. Le lundi 28 mai, vous avez annoncé que le Gouvernement travaillait sur la possible instauration d'une vignette temporelle, afin que les transporteurs routiers contribuent au financement des infrastructures. Cependant, la commission des transports et du tourisme du Parlement européen a adopté, le 24 mai, le rapport de Mme Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy sur la proposition de révision de la directive Eurovignette. Il y est proposé, par l'amendement n° 38, que, à partir du 1 janvier 2021, les autoroutes concédées soient soumises à une redevance pour coûts externes. Il s'agit donc de supprimer progressivement l'utilisation des droits d'usage fondés sur la durée pour instaurer un système basé sur une distance parcourue. Dans ces conditions et si le rapport est définitivement pris en compte, les États membres n'auront plus le choix. Aussi, je vous demande, madame la ministre, alors que vous comptez instaurer un système de vignette pour financer les travaux d'infrastructures et que l'Union européenne semble avoir une autre orientation,

-et, encore plus, à celle des Pays-Bas- 43 % -, de l'Allemagne- 15 % -et de la Belgique- 12 %. Sur 18 000 kilomètres de voies d'eau, la France possède 8 500 kilomètres de voies navigables mais seulement 1 700 kilomètres au gabarit européen. Un maillage fluvial du territoire français existe donc, mais il souffre d'une absence d'interconnexions entre les bassins à grand gabarit. J'y reviendrai plus tard, avec un exemple précis. À cela s'ajoutent les sous-investissements du passé, qui ont aggravé le poids de certains handicaps, entraînant une lente obsolescence de l'infrastructure et laissant notre réseau dans un état d'inadaptation aux conditions d'une nouvelle dynamique du secteur. La France subit ainsi ce déficit fluvial, qui est également la conséquence du défaut d'une stratégie assez globale des pouvoirs publics. Cela a été largement rappelé lors de nos débats, les investissements en faveur des voies navigables demeurent insuffisants dans notre pays. Les investissements actuellement consentis à cette fin, à hauteur de 150 millions d'euros par an, ne permettent pas de maintenir le réseau en état et d'empêcher son vieillissement. Ainsi, certains ouvrages, notamment sur le petit gabarit, se dégradent et deviennent moins fiables, au point qu'il n'est plus possible d'y circuler- c'est le cas, par exemple, Pour les remettre à niveau, nous le savons, il faudrait notamment procéder à des drainages, régénérer les écluses, renforcer l'automatisation et améliorer la sécurité des installations.

II ne faut pas perdre de vue que l'amélioration de notre performance environnementale passe par l'utilisation d'autres modes complémentaires, comme le transport fluvial. Cela a été dit, celui-ci consomme trois fois moins d'énergie que le transport routier. Ce mode de transport dispose de fortes réserves de capacité et peut absorber un important trafic de marchandises. Présent au coeur des plus grandes agglomérations, il offre des itinéraires de contournement des points de saturation, tout en assurant une desserte de proximité. Écologique par sa moindre consommation d'énergie et ses faibles niveaux d'émission de polluants et de CO2, économique par sa capacité de tonnage, fiable par la sûreté de ses acheminements et sa ponctualité, la voie d'eau propose des solutions adaptées aux nouvelles exigences en matière de transport. Je souhaite, madame la ministre, vous interroger sur l'avancement des études en cours relatives à la liaison

à travers ce débat, le groupe Les Républicains et moi-même avons souhaité interroger le Gouvernement sur l'urgente nécessité de mener une politique volontariste en faveur du transport fluvial. Nous en